et d'accompagner une société en mouvement qui a profondément évolué au cours des dernières décennies, certainement de la manière la plus accélérée que l'on ait connue dans l'histoire. Cela

lutter contre les fractures territoriales, d'adapter des solutions de logement pour les plus démunis et de fluidifier, dans la mesure du possible, les parcours résidentiels des plus fragiles.

elles a fait ce qu'elle croyait devoir faire au moment où elle était en poste. Nous voulons faciliter et accélérer l'action de ceux qui construisent, rénovent et aménagent, qu'il s'agisse des collectivités locales, des aménageurs, des bailleurs sociaux, des investisseurs, des promoteurs, des entreprises, des artisans, et ce pour essayer d'apporter le meilleur service possible à nos concitoyens, aux habitants de nos territoires. C'est une véritable innovation de rédiger un texte de loi qui n'ajoute pas de contraintes supplémentaires, mais qui, de manière pragmatique, lève des blocages. S'il arrive que nous ayons

de responsables économiques, syndicaux et culturels nous proposent des amendements très intéressants qui, au fil des années,

à des responsables du secteur de la construction, avec lesquels nous entretenons des relations de confiance constructives, que beaucoup de dispositions législatives et réglementaires étaient en fait la conséquence de leurs demandes. Ils ne l'ont pas nié. En réalité, il est beaucoup plus difficile de simplifier que de complexifier, et nous allons nous en rendre compte au cours de ce débat. Comme vous le savez, ce projet de loi est le fruit d'une large concertation lancée depuis plusieurs mois. Une importante consultation en ligne a été conduite par le ministère et a donné lieu à plusieurs milliers de contributions.

attentif- pour ne pas dire minutieux -par la commission des affaires économiques du Sénat, le texte dont nous allons débattre dans cet hémicycle compte 235 articles, dont les trois quarts sont d'origine parlementaire,

Comme je l'ai déjà dit à vos collègues députés, il serait malvenu de ma part de contester la procédure parlementaire et, plus encore, le droit d'amendement, ... Bravo ! ...

je crois fondamentalement à la démocratie parlementaire, au bicamérisme et à l'importance du travail réalisé ici. Notre état d'esprit est très clair à l'écoute, sans pour autant renoncer, vous le comprendrez, aux principes fondamentaux et aux objectifs premiers de ce projet de loi, qui sont la simplification des procédures et la protection des Français.

objectif de construire plus, mieux et, si possible, moins cher. Il s'agit de libérer et de faciliter les initiatives dans les territoires, en articulant plusieurs leviers.

les collectivités et divers partenaires. Le projet partenarial d'aménagement, le PPA, permettra, par exemple, d'assurer la reconversion d'une ancienne caserne désaffectée pour l'intégrer dans un large projet de rénovation prévoyant logements, commerces, équipements et services. La libération du foncier public sera facilitée grâce à la cession par l'État du foncier de son domaine privé aux signataires d'un PPA.

L'esprit de ces mesures est bien de simplifier, de faciliter, de se retrouver entre partenaires qui ont envie d'avancer et de construire la ville autour d'un projet commun. C'est pourquoi

propos médiatiques que j'ai pu entendre, le texte que je vous présente préserve très largement l'autonomie, l'indépendance et la responsabilité des maires. Dans cette

nous n'avons pas voulu aller au-delà en ce qui concerne le transfert aux intercommunalités. À mon sens, nous avons retenu une solution équilibrée. nous le savons, mesdames, messieurs les sénateurs, l'immense majorité des projets seront coconstruits de façon très apaisée, parce que ces instruments ne seront lancés qu'à la demande des collectivités, et non de l'État. Je le répète, ce sera à la demande des collectivités, pour faciliter et accélérer les procédures et permettre aux grandes opérations

font de la préinstruction en amont pour signifier aux constructeurs qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout de ce que permet le PLU. C'est aussi une réalité de terrain. J'entends, et j'en suis convaincu, qu'il faut défendre et préserver la responsabilité

Autre levier pour faciliter la construction : la simplification des documents d'urbanisme. Si nous allons, comme le souhait en est partagé, vers la simplification, avec une procédure d'instruction dématérialisée

avons ainsi amélioré le cadre législatif actuel en conciliant la préservation du patrimoine littoral, auquel nous sommes tous très attachés, et la réalité économique de nos territoires. Votre commission a déjà apporté quelques évolutions, dont nous débattrons. C'est un sujet sur débattrons. C'est un sujet sur lequel nous ne devons pas être très éloignés. Je n'ai pas de difficultés, par exemple, à prévoir de façon plus explicite des dérogations sur la question des cultures marines pour régler les incertitudes autour de la production conchylicole, mais je veux le réaffirmer très clairement ici : il n'est pas question de revenir sur les règles fondamentales de la loi Littoral, qui est indispensable à la préservation de la biodiversité et du paysage de nos côtes. Elle s'inscrit d'ailleurs pleinement dans le cadre du plan Biodiversité que le Gouvernement a présenté voilà quelques semaines. Ce n'est pas pour rien que j'ai pu envoyer, à la suite des débats à l'Assemblée nationale, un communiqué commun avec Nicolas Hulot sur ce thème. Autre sujet : la simplification des normes de construction pour permettre, par exemple, l'utilisation de nouveaux matériaux, notamment biosourcés, ou encore le développement de logements « évolutifs pour un meilleur équilibre entre adaptation aux besoins de la société, coût de construction et confort des occupants. Là encore, j'entends les interrogations sur le thème de l'accessibilité. Nous en avons largement débattu depuis la loi de 2005 dans cet hémicycle,

leur permettant d'adapter plus facilement leur environnement aux événements de la vie, plutôt que d'appliquer à tous un même cadre rigoureux et mal adapté.

lorsque l'on habite à R+1, R+2 ou R+3, la question de l'accessibilité du logement ne se pose pas, parce que l'on n'y accède pas, le plus souvent. Il faut donc revenir aux fondamentaux

dans nombre d'agglomérations, ce qui est très attendu. Aujourd'hui, on estime à 30 000 le nombre de logements dont la construction est bloquée en France par des recours. Un maire d'une métropole du sud-ouest m'indiquait récemment que 60 % des permis de construire dans sa ville étaient frappés d'un recours. C'est une réalité à laquelle il faut mettre fin ! Comment ?

L'objectif est de rendre ces avis simples pour les installations nécessaires au déploiement de la téléphonie mobile et les opérations de résorption de l'habitat indigne. Ce n'est pas une révolution

Nous proposons enfin, dans le cadre de ces évolutions, un élargissement de la procédure de réquisition des locaux vacants depuis plus d'un an à des fins d'hébergement.

dans tous les domaines, mais particulièrement dans celui-ci -, je puis vous dire qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions ou de tentatives d'évolution qui étaient encore plus frappantes. Il est bien normal que, chaque fois que l'on propose une évolution qui, parfois, est vécue comme une révolution, des résistances se fassent jour. Nous savons ce qu'il en est pour les niches fiscales, mais c'est vrai dans tous les domaines.

Le lien avec les territoires est ainsi garanti, ce qui est pour moi essentiel. Je précise de nouveau qu'il s'agit non pas de contraindre les opérateurs à fusionner, sauf dans le cadre de la même intercommunalité, ce qui concerne un nombre très limité de cas, ni de faire disparaître la diversité des organismes d'HLM ou de leur faire perdre leur identité, mais seulement de fixer l'objectif et de leur fournir une boîte à outils complète pour y arriver. Ce que nous avons fait avec la fédération des des SCOP, chère à Marie-Noëlle Lienemann, ou avec la fédération des EPL, en est la stricte démonstration. Les travaux à l'Assemblée nationale ont permis de mieux prendre en compte certaines dimensions opérationnelles et d'en simplifier la mise en oeuvre. Je pense, par exemple, à la réalité des situations des activités des bailleurs sociaux, notamment des entreprises publiques locales, pour lesquels des règles adaptées ont été définies. Vous avez, là aussi, apporté une modification substantielle en abaissant le seuil de regroupement de 15 000 à 10 000 logements. Je comprends vos interrogations par rapport à cette évolution du secteur- j'ai bien dit « je ». Nous aurions pu obliger les bailleurs à fusionner pour devenir de grands acteurs régionaux, voire nationaux : tel n'est pas notre projet Il faut que, collectivement, nous gardions bien à l'esprit que l'objectif est d'aider les organismes à se renforcer mutuellement, tout en conservant leur diversité. Il n'y a aucun doute à avoir sur ce point. C'est la condition du maintien d'un système du logement social français fort. Or des sociétés de coordination trop petites à l'échelle des territoires ne pourront pas jouer le rôle qui est attendu d'elles. Il faut qu'elles puissent s'arrimer à des organismes de taille intermédiaire. ailleurs, nous souhaitons la simplification du cadre juridique applicable aux bailleurs sociaux, avec de nouvelles mesures pour rendre leur maîtrise d'ouvrage plus efficace C'est d'ailleurs à la demande expresse des bailleurs sociaux que nous avons proposé ces mesures. J'observe notamment que de plus en plus de bailleurs sociaux ont recours aux VEFA avec la promotion privée, car ils ne luttent plus à armes égales quand ils sont en compétition sur le foncier.

Je le dis très clairement, c'est un objectif sur lequel nous n'entendons pas revenir. J'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer à M. le rapporteur pour avis. simplifier l'accession à la propriété pour les locataires d'HLM avec un double objectif simple : d'une part, permettre à des locataires d'acquérir leur logement quand ils le peuvent et le souhaitent et, d'autre part, soutenir la construction ou la rénovation de logements sociaux neufs par les bailleurs. J'ajoute que c'est aussi une solution pragmatique pour stabiliser les classes moyennes dans certains quartiers où la mixité sociale est un enjeu réel. À ce titre, et même si je considère qu'il faut effectivement pouvoir prendre en compte encore plus finement les enjeux des territoires- je l'ai déjà exprimé en séance à l'Assemblée nationale -, je ne suis pas favorable à l'ajout d'une contrainte, avec cet avis conforme du maire pour l'autorisation des ventes d'HLM.

en soi. La nouveauté, c'est de permettre que les objectifs, y compris ceux fixés par les bailleurs sociaux, soient tenus. En troisième lieu, le projet loi cherche à répondre aux nombreux besoins de nos concitoyens en matière de logements et à favoriser la mixité sociale.

grâce à la généralisation de la cotation dans les grandes agglomérations, ce qui ne me paraît pas poser de gros problèmes, et de renforcer la mobilité des locataires dans le parc social en réexaminant tous les trois ans leur situation.

! Nous verrons comment le débat se passe ici. Je souhaiterais également vous dire dès aujourd'hui que je ne suis pas favorable

Je ne pense pas que cela soit une bonne chose. Concernant le parc privé, nous entendons agir avec la création du bail mobilité, contrat de location de un à dix mois non renouvelable et sans dépôt de garantie pour les logements meublés. Il permettra de répondre concrètement aux besoins de personnes en mobilité, étudiants ou travailleurs en mission professionnelle pour une courte durée. J'ai vu d'ailleurs que des amendements intéressants avaient été déposés sur le sujet. Il s'agit là encore

à des loyers abordables pour permettre à des locataires de sortir du parc social. Il s'agit simplement de remettre de la fluidité, de permettre la création de parcours résidentiels. Nous avons aussi la volonté, qui est largement partagée, de favoriser la mixité intergénérationnelle, de plus en plus plébiscitée. Nous avons ainsi prévu une disposition pour sécuriser les aides au logement en cas de cohabitation intergénérationnelle. S'agissant de la colocation dans le parc social, les débats à l'Assemblée nationale ont permis l'adoption d'un amendement tendant à élargir la colocation pour personnes handicapées à une mesure de portée plus générale. d'améliorer les procédures existantes, par exemple en coordonnant mieux celles relatives à l'expulsion et au surendettement pour la colocation.

qui sont mises à exécution. Plus on interviendra en amont, moins il y aura de difficultés ensuite. Nous devons arriver à articuler la procédure devant les tribunaux d'instance et la procédure de surendettement, car il n'est pas sain qu'elles vivent leur vie de manière indépendante l'une et l'autre. Enfin, le texte permettra aux territoires de mieux réguler l'activité, parfois problématique, de la location meublée touristique- tout le monde connaît Airbnb, mais ce n'est pas la seule plateforme. Si cette activité est souvent très utile pour le pouvoir d'achat des Français et l'attractivité touristique de nos régions, dans certaines villes, le marché locatif privé en est trop fortement impacté, au détriment de ceux qui cherchent à se loger.

sénateurs, il y a le sujet SRU. Je veux rappeler ici que le projet de loi ÉLAN n'entend pas toucher aux fondamentaux de la loi SRU, qui a fait la preuve de son efficacité au cours des ans.

Si, à l'Assemblée nationale, une large majorité de députés n'a pas souhaité modifier sur cette question le texte du Gouvernement, à l'inverse, votre commission a adopté de nombreuses évolutions, certaines avec une portée plutôt limitée,

Je reconnais que vos amendements s'appuient sur un certain nombre de situations concrètes que nous connaissons bien. Si le Sénat devait faire évoluer la loi SRU, je ne doute pas, et je le souhaite, qu'il trouvera aussi un équilibre raisonnable, empreint de sagesse. Le président du Sénat, avec sa sagesse légendaire- vous savez l'estime que je lui porte -, a certainement raison lorsqu'il dit qu'« il faut toucher à la Constitution d'une main tremblante ».

Les mesures du projet de loi ÉLAN visent aussi à accélérer la rénovation des centres-villes à travers un contrat intégrateur unique : l'opération de revitalisation des territoires, l'ORT. C'est l'un des objectifs du programme « Action coeur de ville », que j'ai lancé voilà quelques mois pour 222 villes et intercommunalités réparties sur tout le territoire hexagonal et outre-mer, et dont les conventions commencent à être signées par l'ensemble des acteurs- elles seront toutes signées d'ici au 30 septembre.

plus largement à toutes les collectivités qui souhaitent s'emparer d'un outil opérationnel de revitalisation de leur centre-ville. Ce point doit être bien intégré. La liste n'est donc pas bloquée à 222 villes. Je suis également ouvert à la discussion sur la question de l'aménagement commercial dans les villes moyennes, qui fait l'objet d'un certain nombre d'amendements. Comme je vous l'avais dit à l'occasion de l'examen de la proposition de loi sénatoriale adoptée récemment sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, l'examen du présent projet de loi doit permettre de répondre à certaines de vos interrogations et satisfaire nombre de vos préoccupations. Je citerai à cet égard

Nous nous attaquons frontalement à la racine de ce fléau. Il est ainsi prévu d'instituer une présomption de revenus pour les marchands de sommeil comme pour les trafiquants de drogue ; ils seront Le projet de loi systématise aussi les astreintes administratives en cas de travaux prescrits, pour accentuer la pression sur les propriétaires. De plus, en cas d'expropriation, l'indemnité liée sera saisie

Ont été ensuite rendues obligatoires les peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil et d'interdiction d'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de dix ans, sauf décision contraire motivée du juge.

avec eux -, les députés ont adopté une mesure prévoyant que les marchands de sommeil condamnés ne pourront notamment pas acquérir de biens immobiliers en cas de vente par adjudication.

Les amendements adoptés par votre commission sont intéressants. Dans l'esprit de coconstruction qui est le nôtre, ils sont directement versés aux travaux en cours, animés par la Chancellerie et le Gouvernement.

d'y parvenir. Si le Gouvernement maintient sa position initiale, je prendrai devant vous des engagements sur la méthode que nous pourrons adopter pour que le Sénat soit directement et constamment associé à cette évolution. Nous aurons également des discussions autour de la question majeure

Je conclurai sur le numérique, sujet qu'a particulièrement porté, avec talent et conviction, M. le secrétaire d'État Julien Denormandie. Le projet de loi comporte un volet lié aux simplifications dans le déploiement du numérique au profit de tous les territoires. Vous le savez, l'accès à la téléphonie mobile et à une connexion internet de qualité est une attente forte de nos concitoyens et nécessite le déploiement de nouvelles infrastructures. Or le délai moyen d'installation d'un pylône ou d'une antenne est en France de très supérieur à tout ce que l'on constate chez nos voisins européens. Une partie de ces délais est imputable à la réglementation et aux procédures imposées aux opérateurs. Nous avons obtenu d'eux un effort d'accélération inédit, puisque chaque opérateur s'est engagé, sous peine de sanctions, à déployer des milliers de pylônes supplémentaires à ses frais, dont 5 000 pour apporter la téléphonie mobile là où elle est actuellement absente ou insuffisante. des mesures de simplification qui vous sont proposées, nous avons veillé à ce qu'elles permettent l'accélération de ces installations, parfois pour une durée limitée à celle de l'accord, tout en respectant le droit légitime à l'information des maires et des habitants des communes concernées. Je ne doute pas, là encore, que nos débats viendront enrichir le texte actuel en veillant à préserver cet équilibre indispensable entre le désenclavement numérique de nos territoires,

de ce qui a pu être voté et mis en application sous les précédents gouvernements. Nous avons essayé de tirer le bilan

Si le diagnostic posé sur la crise du logement est bon, le texte n'apporte pas toutes les réponses appropriées, qui plus est dans un contexte qui voit toute la chaîne de production du logement neuf ralentir : ventes, mises en vente et mises en chantier sont en net retrait au premier trimestre de 2018 par rapport à la même période en 2017. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, le choc de l'offre a disparu de vos éléments de langage ! Le projet de loi est clairement travaillé par une valse-hésitation constante entre décentralisation et recentralisation. Deux visions antagonistes le portent, au risque de conduire à un produit hybride fait de compromis multiples et d'incohérences absolues. Monsieur le secrétaire d'État, lorsque vous êtes venu devant la commission des affaires économiques, vous nous aviez assurés de votre engagement de coconstruction du texte et que vous étiez ouvert, avec M. le ministre, à toute modification ou tout autre aménagement. Mais il faut croire que votre volonté s'est sérieusement émoussée au regard des amendements déposés par le Gouvernement sur le texte qui reviennent sur les apports du Sénat. Pourtant, la commission des affaires économiques s'est attachée à en corriger les imperfections et à l'enrichir de dispositifs qu'elle a jugés essentiels à la mise en oeuvre d'une politique en matière d'habitat, en s'appuyant notamment sur les conclusions de la conférence de consensus sur le logement. Elle a été particulièrement attentive à la place des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre des politiques locales de l'habitat et, plus spécialement, au rôle des maires. Elle s'est opposée à la recentralisation des dispositifs au profit de l'État, car il existe encore trop souvent des injonctions nationales et des pratiques descendantes très éloignées des préoccupations et des besoins des territoires. Les opérations d'aménagement d'ampleur ne peuvent se réaliser sans les communes. Dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme prévues par des projets partenariaux d'aménagement, la commission a réintroduit l'accord des maires. contre le phénomène de vacance de locaux, la commission s'est attachée à encourager les initiatives locales. Ainsi, elle a prolongé jusqu'en 2023 le dispositif volontaire et contractuel de mise à disposition de locaux vacants par leurs propriétaires en vue de la création de places de logement temporaire. La priorité doit rester le logement ! Dans cette optique, la commission a mieux encadré les conditions de réquisition des locaux à des fins d'hébergement d'urgence, dans le respect du droit de propriété. En ce qui concerne la procédure d'avis des architectes des Bâtiments de France, la commission a considéré que le texte issu de l'Assemblée nationale offrait un consensus équilibré au service de la couverture numérique du territoire et de lutte contre l'habitat indigne. Le Sénat, vous le savez, se fait depuis longtemps le relais du besoin d'adaptation des règles de constructibilité en zones littorale et agricole. Dans la lignée de la proposition de loi de loi de Michel Vaspart relative au développement durable des territoires littoraux et de celle de Jacques Genest visant à relancer la construction en milieu rural, la commission a poursuivi la territorialisation des prescriptions de la loi Littoral et l'assouplissement de la de la règle d'inconstructibilité des zones non urbanisées. Ces mesures faciliteront notamment l'implantation d'annexes, d'équipements collectifs et d'activités de cultures marines. Ce sont des enjeux d'une importance centrale pour le développement démographique, touristique et économique de nos territoires ruraux et littoraux. Le volet relatif à la réorganisation du secteur social n'est que la conséquence des mesures budgétaires de l'automne dernier prises brutalement et unilatéralement, qui ont mis plus qu'à la diète le secteur HLM. Nombre de mesures ne sont que de l'habillage ouvrant à terme la porte à des capitaux privés avec le risque d'une hausse des loyers et l'éviction des plus modestes. Pour autant, la commission n'a pas souhaité remettre en cause les dispositions relatives à la restructuration du secteur social, dont chacun a admis la nécessité. En revanche, elle a apporté des modifications dans sa mise en oeuvre en abaissant les seuils en deçà desquels le regroupement de bailleurs sociaux est obligatoire à 10 000 logements gérés et à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces seuils nous ont paru plus en adéquation avec la situation des bailleurs. Elle a également clarifié les règles d'appartenance à un groupe de logement social, interdisant la double appartenance simultanée à deux groupes d'organismes de logement social. Il nous a paru incohérent de placer les organismes dans des situations insolubles où ils devraient choisir entre les orientations incompatibles de leurs groupes de rattachement. La vente de 40 000 logements sociaux voulue par le Gouvernement est quasi impossible à atteindre, tout le monde, sauf le Gouvernement, le reconnaît. La commission n'est pas opposée à la vente des logements sociaux, mais pas à n'importe quelles conditions. Le maire ne peut pas être laissé de côté. On ne peut pas lui demander de construire plus de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU et, dans le même temps, ne pas lui donner les moyens d'atteindre cet objectif. Nous avons donc prévu son vote conforme sur la vente de logements sociaux. La loi SRU est effectivement la grande absente du projet de loi, puisque seul l'article 46 prévoit d'allonger le décompte des logements sociaux vendus de cinq à dix ans. La commission a adopté plusieurs mesures pour faciliter l'atteinte des objectifs de construction de logements sociaux. Le calendrier actuel est intenable. Si les obligations de la loi SRU ont bien impulsé la dynamique recherchée, l'application uniforme de ce dispositif centralisé apparaît aujourd'hui comme un frein. Combien de temps, messieurs les ministres, allez-vous fermer les yeux sur cette réalité ? La commission a décidé de prolonger les obligations de réalisation de logements sociaux de 2025 à 2031, ce desserrement devant permettre aux communes de réaliser la construction de logements sociaux à un rythme plus soutenable tout en maintenant l'objectif de 25 %. Un calendrier de rattrapage spécifique a été instauré pour les communes « entrantes », les communes nouvelles, qui bénéficieront ainsi de la même durée que les communes actuelles pour réaliser leurs objectifs de construction de logements sociaux. Une expérimentation a été proposée avec la mise en place d'un contrat d'objectifs et de moyens. La liste des logements sociaux décomptés a été complétée de façon restreinte par l'ajout des logements occupés par un titulaire d'un PSLA, des logements objets d'un bail réel solidaire et des places d'hébergement d'urgence. Ces mesures pragmatiques et réalistes permettront aux maires de respecter leurs obligations de construction de logements sociaux dans de bonnes conditions, sans les décourager,

notamment en facilitant la délivrance du congé en cas d'acquisition d'un logement occupé, ou encore en unifiant à deux mois le délai de préavis donné par un locataire, sauf lorsque l'état de santé ou la situation économique du locataire le justifie. La copropriété est un sujet qui touche au quotidien de nos concitoyens. Il ne peut être traité une habilitation à légiférer par ordonnances. La commission a donc adopté plusieurs mesures modifiant les règles de copropriété qui permettront une première amélioration de son fonctionnement. Les squats de logements se développent, vous le savez. Nous ne pouvons rester indifférents. C'est pourquoi nous avons renforcé de nouveau le dispositif de lutte contre les squatteurs, trois ans après l'examen de la proposition de loi sénatoriale tendant à préciser l'infraction de violation de domicile, en prévoyant que les locaux à usage d'habitation bénéficieront des mêmes mesures de protection que le domicile des personnes. La commission a également contribué au renforcement de l'efficacité du dispositif de lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Nous avons rendu plus efficaces les permis de louer et de diviser en donnant au maire l'accès au casier judiciaire des demandeurs. Nous avons étendu aux agents immobiliers l'obligation de déclarer au procureur de la République les suspicions d'activités de « marchands de sommeil ». Considérant qu'une ligne rouge avait été franchie, la commission a enfin supprimé deux points de l'ordonnance relative aux polices de lutte contre l'habitat indigne. S'agissant des dispositions destinées à assurer la revitalisation

au déploiement des réseaux numériques, la commission a souhaité, avec la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, aller plus loin que le projet de loi issu de l'Assemblée nationale afin de répondre aux attentes de nos concitoyens en la matière, sans pour autant priver les maires de leurs prérogatives. Elle a notamment répondu à une forte demande des élus de montagne comme des opérateurs, en insérant explicitement dans la loi une dérogation au principe de construction en continuité d'urbanisme en zone de montagne. Elle a également entendu crédibiliser les engagements des opérateurs en renforçant les sanctions encourues en cas de manquement à ces engagements et en étendant leur champ d'application. Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le texte tel que la commission l'a modifié. La parole est à M.

que le projet de loi ÉLAN comporte un certain nombre de dispositions visant à simplifier les normes et les procédures d'urbanisme. Parmi ces règles auxquelles le projet de loi apporte des modifications, ou qu'il prévoit d'assouplir, figurent plusieurs dispositions destinées

Face à l'ampleur de la crise du logement que connaît notre pays, je comprends parfaitement le souhait de vouloir donner aux entreprises et aux acteurs les capacités d'inventer des solutions nouvelles, de réduire les délais de production de logements, de construire et de rénover davantage. Faut-il pour Faut-il pour autant prendre le risque de remettre en cause la qualité architecturale et la mise en valeur du patrimoine, deux éléments pourtant indispensables à l'attractivité de nos territoires et à la qualité de vie ? tant nous sommes tiraillés entre plusieurs objectifs d'intérêt général, aussi louables les uns que les autres, mais qui entrent en contradiction entre eux. Le débat n'est pas nouveau. En 1962, lorsqu'il a présenté devant le Parlement le projet de loi qui allait porter son nom, André Malraux pointait déjà du doigt ce paradoxe, évoquant la nécessité « de concilier deux impératifs qui peuvent paraître opposés conserver notre patrimoine architectural et historique et améliorer les conditions de vie [ ...] des Français ». Exactement ! Alors même que la situation en matière de logement était plus tendue encore à l'époque qu'aujourd'hui, c'était la volonté de trouver le point d'équilibre entre ces différents principes apparemment contraires qui animait André Malraux. Tel n'est malheureusement pas l'objectif du projet de loi ÉLAN, qui semble davantage faire primer la construction de logements sur toute autre considération d'intérêt général, comme le laisse à penser l'étude d'impact. C'est vrai ! Or le risque de cette orientation, c'est de nous faire répéter les erreurs d'urbanisme d'après-guerre, dont nous payons encore aujourd'hui le prix.

de remettre en cause. L'instabilité juridique que le projet de loi pourrait générer soulève d'autant plus d'inquiétudes qu'elle intervient dans des domaines où la stabilité des normes est particulièrement importante. La préservation du patrimoine est une action qui s'inscrit dans la durée et s'accommode mal des règles mouvantes.

Je sais qu'il souffre d'une image de fonctionnaire parfois « buté » en dépit du faible nombre de refus qu'il oppose chaque année et des possibilités de recours qui existent contre ses décisions, à l'occasion desquelles les commissions régionales du patrimoine et de l'architecture, présidées par des élus, sont désormais consultées. Le but de l'avis conforme- dois-je le rappeler ? -est de garantir que les enjeux patrimoniaux puissent aussi être pris en compte, au même titre que d'autres enjeux. Ne nous y trompons pas, les quatre cas qui nous sont soumis aujourd'hui sont loin d'être anodins et pourraient entraîner des atteintes irréversibles à notre patrimoine. Renoncer à l'avis conforme privera certes l'ABF de sa capacité d'empêcher un projet, mais lui retirera également toute possibilité d'établir un dialogue pour permettre qu'un projet évolue dans le sens d'une meilleure conciliation de tous les intérêts en présence. La commission de la culture vous proposera quelques amendements allant dans le sens d'une plus grande coconstruction des projets entre les élus et les ABF et d'une meilleure prévisibilité des avis de ces derniers. Voulons-nous vraiment prendre le risque que le maire soit désormais seul et sans protection face à la pression des promoteurs de projet pour décider ? Voulons-nous vraiment ouvrir une brèche au principe de l'avis conforme pour que la liste des exceptions ne fasse que s'allonger au fil des années, au point de le vider de son sens ? Compte tenu de l'atout que représente le patrimoine pour notre pays et ses territoires, ce serait, aux yeux de la commission de la culture, une erreur. La parole

la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est saisie pour avis de vingt-sept articles du projet de loi que nous examinons aujourd'hui : onze sont relatifs à l'aménagement numérique du territoire, trois ont trait qui prolongent les travaux effectués par la commission sur ce sujet depuis plus de cinq ans, et treize touchent à des sujets plus ponctuels concernant l'évaluation environnementale, la participation du public, la qualité de l'air intérieur ou encore l'eau et l'assainissement. Avec ce périmètre de saisine large et des délais d'examen très contraints du texte au Sénat, la commission a fait le choix de concentrer son avis sur deux sujets au coeur de ses compétences le volet « numérique », vous vous en doutiez, et, sur l'initiative de notre collègue Michel Vaspart, président du groupe d'études Mer et littoral, les dispositions relatives, non pas à la loi Littoral, mais à des mesures pragmatiques concernant le littoral. Au-delà de ces éléments liminaires, je souhaite partager avec vous un constat sur la méthode : le projet de loi ÉLAN est devenu un monstre législatif. Monsieur le ministre, que la diversité des sujets abordés, sans réelle cohérence d'ensemble, ne permet pas aux commissions permanentes compétentes du Parlement de travailler correctement. Au-delà de l'objectif de simplification, qui devrait d'ailleurs être considéré davantage comme un moyen que comme une fin en soi, l'objet du projet de loi ÉLAN est devenu difficile à cerner, ce qui nuit à la qualité du travail parlementaire. En outre, si l'ambition affichée par le Gouvernement est grande, elle ne concerne pas tous les aspects du texte dans la même mesure. Je tiens, à cet égard, à vous témoigner ma déception à propos de la pauvreté de la partie « N » du projet de loi consacrée au numérique, qui comportait seulement quatre articles dans le projet de loi initial, sur soixante-cinq. Les discussions qui ont eu lieu sur le sujet à l'Assemblée nationale n'ont pas permis de rééquilibrer cette asymétrie, et les mesures proposées me paraissent très en deçà des besoins des acteurs du secteur. De nombreuses lacunes demeurent, que ce soit sur la mutualisation des réseaux, le contrôle des obligations de déploiement des opérateurs ou encore sur l'évaluation de la qualité de la couverture mobile proposée à nos concitoyens.

Nous abordions aussi ces thèmes dans le rapport d'information sur le très haut débit pour tous en 2022, adopté par la commission en 2017 et que nous avons élaboré avec le président Hervé Maurey.

La commission a adopté dix-huit amendements, dont seize sont intégrés au texte que nous examinons aujourd'hui. Sur l'initiative de notre collègue Michel Vaspart, nous avons souhaité rendre plus opérationnelles les dispositions votées à l'Assemblée nationale concernant le littoral, en particulier sur le sujet des dents creuses dans les communes littorales, avec, comme je l'ai déjà dit, des propositions équilibrées et pragmatiques. La commission a également souhaité renforcer le volet relatif à l'aménagement numérique du territoire avec deux objectifs d'une part, l'accélération des déploiements des réseaux en fibre optique ; d'autre part, l'amélioration de la couverture mobile. Il faut mieux associer les collectivités territoriales pour assurer le respect des engagements souscrits par les opérateurs, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, améliorer la transparence de l'information nécessaire au déploiement et organiser efficacement le marché des services de communications électroniques. Nous l'avons vu encore hier, c'est en jouant collectivement que l'on peut gagner. C'est le sens des modifications apportées au texte de l'Assemblée nationale et des cinq articles additionnels insérés sur l'initiative de notre commission au sein du chapitre VI du titre IV portant sur l'amélioration du cadre de vie, qui doit contribuer à apporter à tous les Français un accès de qualité aux techniques et aux usages numériques. C'est, je crois, un élément central de la cohésion territoriale et une nécessité économique. Sous le bénéfice de ces observations, la commission vous propose, mes chers collègues, d'adopter les articles dont elle est saisie.

d'ici à la fin de l'année et qui marque le début de cette crise de confiance après les annonces fiscales et financières qu'a faites le Gouvernement l'an dernier. Tous les indicateurs nous laissent à penser que nous allons connaître dans les deux ans qui viennent non pas un choc de l'offre, mais un choc sur l'offre de logements. Plusieurs gouvernements ont tenté de combattre cette fameuse crise du logement, due à des problèmes essentiellement démographiques. Ceux qui y ont réussi partiellement le doivent souvent à des questions de méthode. Ce fut le cas pour la loi de cohésion sociale, présentée il y a quelques années par Jean-Louis Borloo, dans un contexte de chômage aussi important qu'aujourd'hui, qui a permis d'augmenter de 50 % le nombre des constructions et de tripler le financement du logement social. Ce fut le cas également lorsque Mme Pinel proposa des mesures pragmatiques de relance du logement. Il n'y a donc pas de fatalité à la crise du logement.

dans les textes et les prises de position du Gouvernement. Le président Larcher l'a dit : il faut adopter une approche pragmatique qui prenne mieux en compte les besoins et les spécificités des contraintes de tous les territoires, et il y a urgence à simplifier les nouveaux dispositifs. Force est de constater que le projet de loi n'est pas un texte de décentralisation- notre excellente rapporteur au fond l'a dit -, puisque, dès ses premiers articles, il prévoit de créer de nouveaux outils outils permettant de dessaisir le maire de ses prérogatives et d'introduire le préfet quasiment à tous les niveaux dans le cas de grandes opérations d'urbanisme, dont l'utilité reste à démontrer après l'échec retentissant des opérations d'intérêt national. Plusieurs autres articles dénotent une méfiance certaine du Gouvernement vis-à-vis des élus locaux, en particulier des maires. Il y a donc une nécessité impérative pour le Sénat de réintroduire le rôle du maire, qui est central dans tout ce qui touche à l'utilisation et à la régulation du droit du sol.

Enfin, ce texte ne s'attaque pas vraiment aux deux contraintes majeures qui contrarient l'augmentation de la construction dans le pays : la contrainte financière, qui a fait l'objet de discussions dans la loi de finances, qui privilégie les zones tendues au détriment

des SCOT, de plus en plus enserrés, obérés par des prescriptions environnementales toujours plus lourdes qui raréfient considérablement le foncier disponible. Certes, on peut faire du renouvellement urbain, mais cela a des limites. Il y a donc une contradiction entre vouloir construire plus et ne pas simplifier ces règles d'urbanisme.

et de simplification. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par nos excellents collègues Dominique Estrosi Sassone, Patrick Chaize et Jean-Pierre Leleux et insisterai sur les aspects majeurs de ce texte nous concernant. Lorsqu'on touche au droit de la copropriété, au pouvoir de police du maire, pour ne prendre que ces exemples, il n'est pas sain, monsieur le ministre, de procéder par ordonnance et de priver ainsi le Parlement de son pouvoir législatif, alors qu'il est le garant de l'équilibre des territoires et des relations entre les propriétaires et les locataires. En outre, nous avons proposé un amendement visant à expérimenter une mutualisation intercommunale- notre collègue Dominique Estrosi Sassone l'a fait pour l'échelle communale -pour atteindre les objectifs de la loi SRU. Il ne s'agit en rien de la détricoter, puisque

En conclusion, je dirai que ce texte comprend plusieurs points positifs pour accélérer la construction, notamment la lutte contre les recours abusifs et la lutte contre l'habitat indigne, mais il manque un ingrédient essentiel- je l'ai dit au début, et j'en termine par là la confiance dans les territoires, la confiance dans les élus locaux, que nous proposons de réintroduire par plusieurs amendements, alors même que plusieurs gouvernements précédents s'étaient appuyés avec succès sur cette confiance pour réussir à résoudre la crise du logement. Mais, c'est vrai, c'était dans l'ancien monde

12 millions de personnes sont fragilisées par rapport au logement, par le surpeuplement, les impayés, l'insalubrité ou la précarité énergétique. Ce sont les chiffres du rapport de la fondation Abbé-Pierre. Rappelons-nous que, derrière ces chiffres, il s'agit quand même de 15 millions de nos concitoyens. Le Président lui-même l'a dit : personne ne peut supporter aujourd'hui, dans notre pays, que des gens dorment et meurent dans la rue. Nous ne supportons pas non plus, pour notre part, que reprenne chaque 1 avril le ballet des expulsions locatives sans relogement pour des personnes toujours plus fragilisées et précarisées, prises dans la spirale infernale du déclassement et de l'exclusion. Cela ne va nullement s'arranger avec votre politique générale. Avec l'emploi, l'éducation et la sécurité, le logement est une priorité de nos concitoyens, du fait de la cherté et du manque de logement. Face à ce défi du mal-logement, qui ronge notre pacte républicain, il faut des réponses fortes, globales et structurantes de la part des pouvoirs publics. À l'inverse, nous avons là un texte qui prône la dérégulation, la déréglementation et la privatisation du patrimoine de la Nation. Sur la forme, nous pouvons regretter un texte lourd, véritable de mesures, sans autre fil directeur que celui du désengagement de l'État de ce secteur d'intérêt général répondant à un droit constitutionnel. De 66 articles initialement, ce texte a triplé à l'Assemblée nationale, et le Sénat ne l'a pas allégé. Il est aujourd'hui plus épais que le code du travail. Il est d'ailleurs à noter que, lorsqu'il s'agit de protéger les salariés, vous trouvez le code du travail trop volumineux, archaïque, alors qu'il est l'héritage d'un siècle de luttes et de conquêtes sociales. En revanche, lorsqu'il s'agit de casser notre modèle du logement unique en Europe en quelques semaines, la complexité n'est étrangement plus un problème insurmontable pour vous, l'épaisseur est même moderne, car elle est l'un des outils au service de votre politique de casse sociale. Monsieur le ministre, reprenons en quelques mots le chemin de croix que va affronter un futur demandeur de logement social. Une fois qu'un demandeur aura accès à un logement- sept ans en moyenne aujourd'hui à Paris -, il lui sera plus difficile de s'y maintenir par la procédure de réexamen de sa situation tous les six ans. Certes, la mobilité ne sera pas imposée, mais il sera facile de faire pression sur les locataires. Pour les jeunes, ce sera le bail mobilité, appelé bail précarité par les associations tellement l'équilibre dans les relations entre bailleurs et locataires sera défavorable. Quel avenir pour ces jeunes qui auront disposé d'un bail mobilité de un à dix mois ? Les enchaîner pendant toutes leurs études ? Retourner chez leurs parents ? Aller engraisser les marchands de sommeil ? Pour les personnes en situation de handicap, ce seront seulement 30 % des nouveaux logements qui seront accessibles au lieu des 100 % prévus actuellement par la loi. Pourquoi ? Pour rogner quelques mètres carrés pour des logements toujours plus petits ? Nous avons déjà perdu dix mètres carrés en dix ans. Par contre, pour les promoteurs et autres bailleurs, c'est Noël avant l'heure. La loi MOP est largement contournée, le concours d'architecture supprimé, la loi Littoral malmenée. L'avis des architectes des Bâtiments de France est rendu simplement consultatif. Pour faire vite, toute entrave à la construction, à la production de béton est levée par ce projet de loi, indépendamment des objectifs environnementaux, de préservation du foncier et de la qualité du bâti. Pourtant, mes chers collègues, le beau, ce doit être aussi pour le logement social, qui a été le lieu de toutes les innovations architecturales. Vous vouliez « construire mieux, plus et moins cher ». En réalité, vous construirez moins, en plus laid, pour enrichir toujours les mêmes ! Monsieur le ministre, le logement, en France, repose sur deux jambes : l'une privée, l'autre publique. Ce modèle est unique en Europe, depuis que Mme Thatcher en a détruit la version anglaise. C'est grâce à cette jambe publique que nous avons pu répondre à l'appel de l'abbé Pierre en 1954, ou encore qu'en 2008, pendant la crise des, près près de 50 000 logements ont été déstockés par les bailleurs sociaux auprès des promoteurs pour qu'ils ne mettent pas la clé sous la porte. Votre projet de loi ampute cette jambe publique. Pourtant, pour marcher, il faut les deux jambes Votre projet de société, c'est la précarité de la naissance à la mort ; votre devise, c'est « la France, une chance pour chacun », comme l'a dit le Président de la République lors de l'enterrement de première classe du plan Borloo. Mais, comme quand on signe un contrat, il ne faut pas oublier de lire les petits caractères en bas une chance pour chacun, oui, surtout, si vous êtes bien né ; pour les autres, ce sera la galère à vie ! Monsieur le ministre, la France est un pays qui a une histoire, et cette histoire se respecte. On peut être de droite ou de gauche, mais on s'inscrit dans cette histoire. Nous avons un modèle social unique, que le monde entier nous envie, héritage de luttes sociales et de compromis entre différentes forces politiques, syndicales et sociales. Nous devons en être fiers On peut vouloir réformer, innover, mais la France a cette histoire singulière et ne se dirigera jamais comme une start-up de la Silicon Valley. Très bien ! En réalité, votre projet de loi apporte sa pierre à un édifice construit depuis les années soixante-dix et les lois Barre de marchandisation du logement. Après la dernière loi de finances, qui a privé les bailleurs sociaux de près de 1,5 milliard d'euros, vous portez le coup de grâce au tissu d'HLM en les obligeant à vendre leur patrimoine, par lots, à la promotion privée. Pour favoriser cette gestion déshumanisée du patrimoine, vous les obligez dans la droite ligne de la loi ALUR à se regrouper, portant une atteinte forte à l'impératif de proximité. nous le savons toutes et tous dans nos territoires, avec les politiques de logement, c'est cette proximité, ce lien avec les populations qui est fondamental. Vous encouragez cette vente par le décompte de ces logements pendant dix ans au titre de la loi SRU, renvoyant aux prochains mandats les nécessaires efforts de construction. Vous supprimez la taxe d'habitation et réduisez les dotations aux collectivités, qui se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité de mener des politiques audacieuses en matière d'habitat. Vous créez les conditions d'une explosion prochaine du mal-logement, en affaiblissant l'offre publique de logement déjà saturée. Près 2 millions de personnes en attendent un aujourd'hui ! Mes chers collègues, le passage en commission au Sénat du projet de loi a permis une avancée et donné lieu à un recul : une avancée sur le rôle des maires, que ce soit en matière d'urbanisme ou d'avis pour la vente des logements sociaux sur leur territoire ; mais un recul majeur, celui du détricotage du détricotage de la loi SRU. Droit dans les yeux, je vous le dis : nous ne vous laisserons pas faire ! Il est usant de devoir rappeler que la loi SRU a permis la construction de plus de 500 000 logements depuis près de vingt ans. Ici, la majorité de droite ne veut pas parler de détricotage, alors elle emploie le mot « expérimentation ». Pourtant, la loi SRU et les obligations qui en découlent doivent être respectées. Nous ne pouvons accepter que certains élus fassent du non-respect de cette loi un argument de campagne politique, souhaitant protéger les ghettos de riches peu excessif ! Dois-je vous rappeler que, suivant le dernier décompte, 1 152 communes étaient concernées et que 649 n'ont pas rempli leur objectif, seulement 269 étant carencées ? On est donc bien loin encore d'avoir atteint les objectifs initiaux L'obligation républicaine de solidarité doit être respectée. La mixité et le partage des espaces sont les conditions du vivre ensemble et d'une société apaisée. apaisée. Nous souhaitons faire des propositions d'avenir pour que le logement public reste le creuset de l'égalité républicaine, l'outil de la réalisation du droit au logement et à la ville. Premièrement : interdire les expulsions sans relogement, pratique barbare, et mettre en place une sécurité sociale du logement pour apporter de la sécurité aux locataires comme aux bailleurs. Deuxièmement : renforcer la régulation des loyers dans le secteur privé comme public. Il faut maintenir l'encadrement des loyers, mais en permettant leur baisse effective. Troisièmement : en finir avec les surloyers qui excluent, en relevant les plafonds d'accès au logement social pour diversifier les publics, et aussi redonner des marges de manoeuvre financières aux organismes d'HLM. Enfin, nous accordons une attention spécifique à la question foncière, obstacle majeur à la construction. Nous proposons la création d'une agence foncière pour le logement, qui serait le support d'un domaine public du logement. L'État, garant du droit au logement, en serait propriétaire, et l'usufruit serait confié aux bailleurs. Ce patrimoine serait inaliénable et aurait vocation à reprendre du terrain sur le secteur marchand. Pour mener ces politiques, nous souhaitons que l'État se réengage dans les aides à la pierre en réorientant l'argent des niches fiscales, qui portent le nom de tous les ministres de la ville successifs et pèsent 2 milliards d'euros dans le budget de l'État et qui sont même contestées par la Cour des comptes. Nous souhaitons que les employeurs contribuent plus encore aux bonnes conditions par un retour du 1 % à son taux initial. Nous voulons enfin que les maires disposent financièrement et en droit de tous les outils leur permettant de répondre à l'urgence sociale. Avant de voter cette motion tendant à opposer la question préalable, méditons sur cette phrase de l'abbé Pierre Chaque fois que l'on refuse 1 milliard pour le logement, c'est 10 milliards que l'on prépare pour les tribunaux, les prisons et les asiles de fous. » La parole

le groupe Les Républicains est contre la motion présentée par les sénateurs du groupe CRCE tendant à opposer la question préalable. Nous partageons certaines remarques et regrettons certains aspects du projet de loi, par exemple le contournement du rôle des maires au profit des intercommunalités. Nous regrettons également que, loin de provoquer un « choc de construction », les premières décisions du Gouvernement en matière de logement ont conduit à l'effet inverse

étant, la commission s'est attachée à corriger le texte initial et à lui redonner du souffle. La commission des affaires économiques a ainsi rétabli le rôle du maire, a apporté des aménagements concernant la restructuration du secteur du logement social et l'attribution de logements, a introduit de nombreux dispositifs concernant la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, a amélioré les conditions d'accessibilité des logements neufs, a renforcé la régulation des meublés de tourisme. Sur la simplification des documents d'urbanisme, de nettes améliorations ont été apportées. Sur le numérique, le texte a également été enrichi pour atteindre les objectifs de couverture du territoire. La commission a également introduit des dispositifs sur des sujets totalement absents du texte, mais pourtant essentiels pour le logement : c'est l'exemple des relations entre bailleurs privés et locataires ou des aménagements nécessaires à la loi SRU pour que les maires atteignent dans de bonnes conditions les 25 % de logements sociaux. Il est donc nécessaire d'examiner le projet de loi et de continuer, à travers nos débats, à l'améliorer, d'autant plus que la conférence de consensus a permis à l'ensemble des acteurs du logement de travailler et d'être associé à ce texte. Quel

intéressant. Bien sûr, la situation politique a évolué depuis un an, mais je me suis bien gardé de faire le procès des gestions antérieures.

en septembre 2017. Le Sénat n'a pas attendu que le texte arrive aux portes du Palais du Luxembourg pour se saisir de la question du logement. Dès l'été 2017, la conférence de consensus, initiée par Gérard Larcher, a invité l'ensemble des acteurs du secteur à se prononcer sur les principaux axes de la réforme la place des collectivités dans la politique du logement, l'accélération de la construction, la simplification normative, la réforme du logement social, la cohésion territoriale et le dynamisme des centres-villes. Par ailleurs, une large majorité de sénateurs a soutenu la proposition de loi initiée par Rémy Pointereau et Martial Bourquin pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Issu d'un long travail de concertation, le texte gouvernemental comptait à l'origine 65 articles ; nous en sommes aujourd'hui à 234, qu'il nous faudra examiner, avec plus de 1 000 amendements, en l'espace de sept jours pour simplifier et libéraliser le secteur du logement. Tout au long des discussions, le groupe Les Indépendants sera particulièrement attentif à l'équilibre qu'il nous faut trouver entre libéralisation du secteur et progrès social et environnemental. À ce titre, notre groupe a porté une disposition, adoptée en commission, qui prévoit de recueillir l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur les dérogations à la loi Littoral. Nous veillerons également à ce que l'autorité des maires soit préservée en matière de politique du logement afin de respecter la diversité locale. Pour faire face à la crise du logement, il s'agit d'abord d'aligner la stratégie de construction sur les besoins des populations et des territoires. À travers ce texte, le Gouvernement entend maintenir le rythme de production de logements pour permettre au parc d'absorber les évolutions démographiques, en particulier dans les zones tendues. Le secteur doit faire face, si l'on y ajoute les demandes locatives et d'acquisition, à une demande d'environ 2,7 millions de logements par an. À cet effet, les grandes opérations d'urbanisme et les contrats de projet partenarial d'aménagement représentent des outils intéressants. Nous saluons la volonté de la commission des affaires économiques du Sénat de maintenir l'avis conforme du maire comme préalable à tout transfert de compétence en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, le texte propose plusieurs dispositifs visant à lutter contre la vacance, qui renchérit le coût des logements. Il entend faciliter la conversion de bureaux en habitations et la mise à disposition de logements vacants, tout en encadrant plus strictement les modalités de réquisition des bâtiments à des fins de logement d'urgence pour préserver le droit de propriété. Ce texte vise également à simplifier les normes applicables en matière de logement. Le Gouvernement a ainsi proposé d'instaurer un gel normatif sur la durée du quinquennat pour la construction, à l'exception du champ de la sécurité. L'une des principales mesures de simplification prévoyait une baisse drastique des taux d'accessibilité dans l'habitat collectif neuf. Nous avions proposé de relever ce taux à 25 % en commission, mais avons été devancés par une proposition de la rapporteur allant dans le même sens. Ces redressements sont importants, non seulement pour favoriser l'inclusion sociale des personnes porteuses d'un handicap, mais aussi pour préparer la société aux conséquences sur le logement du vieillissement de la population. Il s'agit également d'accélérer les procédures de contentieux, nombreuses en matière d'urbanisme. Les règles concernant les autorisations délivrées par les architectes des Bâtiments de France ont également été légèrement remaniées en ce qui concerne l'implantation d'antennes relais et la rénovation d'habitats insalubres ou en ruine. C'est un difficile équilibre qui a été trouvé entre la commission des affaires économiques et la commission de la culture, comme sont parfois- et non pas souvent -difficiles les relations entre maires et ABF. Mais nous savons tous qu'il y a des maires démolisseurs et des ABF butés. Autre dimension du texte : la refonte profonde du secteur des habitations à loyer modéré contribuera à leur équilibre économique. Une nouvelle dynamique devrait voir le jour dans les parcours résidentiels sociaux, avec l'allongement de la durée de décompte dans les quotas de la loi SRU des logements sociaux vendus. En janvier 2017, le taux de mobilité était de 6,8 % en Île-de-France, contre une moyenne nationale de près de 10 %. La baisse de la mobilité résidentielle s'est accentuée, en lien avec la crise économique, en particulier dans les grandes agglomérations. La création d'un bail mobilité devrait contribuer au développement d'une offre de logements adaptés à la diversité des situations vécues. Troisième dimension du texte, l'amélioration du cadre de vie passe par la rénovation des passoires thermiques. Dans le parc ancien, les réhabilitations nécessaires du chauffage ou de l'isolation sont coûteuses, notamment pour les logements datant des années Nous défendrons un amendement visant à valoriser les actions d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments prises de façon pionnière par les acteurs du secteur tertiaire. À travers ces dispositions, le projet de loi est un pas vers l'adaptation de notre politique de logement aux grandes évolutions de la société. Nous espérons qu'il sera, à l'issue des discussions, à la hauteur des attentes de nos concitoyens.

projet de loi porte sur des questions majeures. Le logement est un sujet fondamental pour les Françaises et les Français, pour la cohésion sociale de notre pays.

Pour ce qui concerne la lutte contre les marchands de sommeil, on ne peut que saluer les mesures proposées. De même, pour ce qui concerne la nécessaire transition énergétique, le texte fait un pas dans la bonne direction. Mais, en tant qu'écologistes, nous souhaitons qu'il aille plus loin. Nous ferons, à cette fin, certaines propositions. Sur la question de l'artificialisation des sols, certaines mesures vont dans le bon sens, notamment la réhabilitation des centres-villes, qui permet d'éviter l'étalement urbain. Je souhaiterais néanmoins que le texte soit davantage mis en cohérence avec le récent plan Biodiversité et, notamment, que soit inscrit dans la loi l'objectif « zéro artificialisation nette du territoire en 2025 », annoncé par Nicolas Hulot.

De même, l'aménagement du territoire, la qualité des constructions et celle des paysages sont des enjeux où l'intérêt général ne recoupe pas toujours l'intérêt privé. Sur le modèle du logement social qui est proposé, là encore, nous ne pouvons qu'exprimer certaines inquiétudes. Certes, le fait de réexaminer la situation des locataires tous les trois ans permettra une attribution plus juste des logements. Cependant, les autres mesures du texte posent question. On ne peut que s'interroger sur la vente des HLM, telle qu'elle est proposée par le projet de loi. Le risque est important de diminuer l'offre de logements sociaux, dans un contexte de baisse des recettes des organismes d'HLM. La version de la commission a, quant à elle, été bien plus loin encore. Elle porte atteinte de manière, selon nous, inacceptable à la loi SRU, pourtant essentielle à la mixité sociale et pour l'accès au logement. Sur la question de l'accessibilité, le texte suscite aussi des inquiétudes. Nous proposerons de rendre l'ensemble des logements réellement évolutifs, en installant un ascenseur dans toutes les constructions à étages. Les droits des personnes handicapées et le vieillissement de la population nous imposent de ne pas considérer cette problématique comme un simple surcoût. outre, des garanties doivent être apportées aux locataires, notamment sur le bail mobilité. Nous défendrons également des amendements en ce sens. Enfin, je citerai un enjeu sur lequel il nous faudra, dans un avenir proche, nous pencher sérieusement : celui de l'accueil des migrants. Cet accueil pourrait et devra se faire sur l'ensemble du territoire, notamment dans les communes rurales. Il s'agit là, selon nous, d'une formidable occasion de revitaliser les campagnes,

Le projet de loi ÉLAN est en effet la traduction législative de la stratégie de logement engagée par le Gouvernement. Il est également le fruit de la méthode de La République En Marche : la concertation, l'écoute et le dialogue. depuis mai 2017, vous avez rencontré les élus des territoires, les professionnels, les acteurs associatifs du monde du logement, de l'urbanisme et du numérique. Dans le prolongement de ces premières discussions, une large conférence de consensus s'est tenue ici, sur l'initiative du Sénat avec la bienveillance du Gouvernement. Ces consultations ont permis d'associer à la discussion du texte plus de 20 000 contributions émanant des citoyens, des professionnels du secteur ou même des parlementaires. Cette méthode de concertation et de coconstruction a été saluée par tous. Le dialogue va donc se poursuivre dans notre hémicycle pendant les sept jours à venir. Certaines répétitions générales ont déjà eu lieu cette année. Elles permettront d'enrichir le projet de loi ÉLAN. Je pense notamment à nos débats consacrés à la proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes la proposition de loi de M. Chaize sur les infrastructures numériques ou encore aux diverses propositions de loi relatives au littoral. Le logement est l'une des préoccupations majeures des Français. Nous ne sommes pas ici pour faire une loi de plus sur le logement- il y en a eu précédemment, et j'en ai d'ailleurs examiné plusieurs -, mais pour répondre aux besoins des Français. pouvons-nous nous satisfaire de 4 millions de mal-logés aujourd'hui ? Non ! Pouvons-nous accepter que des familles vivent dans des taudis à des prix indécents ? Non ! Pouvons-nous nous satisfaire que plus de 2 millions de Français attendent encore un logement social ? Non Pouvons-nous accepter que deux jeunes adultes sur trois habitent encore chez leurs parents et renoncent à des opportunités professionnelles parce qu'ils ne trouvent pas de logement ? Non ! Pouvons-nous accepter qu'il y ait toujours, dans notre pays, des zones grises et blanches où les Français ne sont pas connectés au très haut débit ? Non Nous sommes d'accord : une réforme ambitieuse est aujourd'hui nécessaire. Nous devons apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets. C'est dans ce cadre, celui d'une méthodologie éprouvée et d'une réforme ambitieuse, que s'inscrit le projet de loi ÉLAN. vise deux objectifs principaux. Le premier est de protéger afin de donner plus à ceux qui ont moins. Il s'agit de renforcer le modèle du logement social, de favoriser la mobilité dans le parc social et de rendre plus transparentes les attributions de logements par les commissions, de lutter de lutter enfin contre l'habitat indigne. Le second objectif est de libérer pour responsabiliser. Il faut offrir de nouvelles opportunités en facilitant la démarche de construction tout en responsabilisant les acteurs du logement quant aux objectifs à atteindre pour construire et rénover plus de bâtiments. Monsieur le projet de loi ÉLAN s'inscrit dans la volonté de préserver la cohésion entre nos territoires, au coeur de la mission qui vous a été confiée par le Président de la République : donner à toutes et à tous les mêmes chances de réussir et de s'épanouir. C'est en créant de nouvelles solidarités que nous réduirons la fracture territoriale. Les quatre titres du présent projet de loi fixent quatre grandes orientations. Elles ont été largement enrichies par nos collègues députés. La première orientation mieux et moins cher, en donnant aux professionnels les moyens d'être plus efficaces, par exemple à travers la dématérialisation du permis de construire, mais aussi en réduisant l'insécurité juridique liée aux recours contentieux ou à la multiplication des normes. À ce titre, la pause normative prévue sur la durée du quinquennat est une excellente initiative. À force, les surcoûts engendrés par l'inflation normative ont fini par freiner la construction et l'innovation.

en rendant plus transparentes les attributions de logements sociaux, en luttant contre l'habitat indigne et en favorisant la mixité, dans les deux sens : les logements sociaux ne doivent pas devenir des ghettos de pauvres, mais accueillir des gens de niveaux sociaux différents. Répondre aux besoins de chacun, c'est aussi favoriser la mobilité dans le parcours résidentiel et lutter contre l'assignation à résidence. Vous proposez ainsi, monsieur le ministre, de construire plus ; vous proposez de favoriser la mobilité dans le parc d'HLM ; vous proposez la mobilité sociale et professionnelle avec le bail mobilité.

évidemment, achever la couverture numérique de notre territoire. Comme nous pouvions le prévoir, le texte a été profondément modifié lors de son examen en commission. Madame la rapporteur, vous avez suggéré de nombreuses évolutions, pas toujours dans le sens que nous souhaitions.

clause pénale qu'avait supprimée la loi ALUR, et nous nous opposons à la suppression des délais de délivrance du congé donné au locataire en cas de vente. Ensuite, en matière d'attribution de logements sociaux, nous souhaitons maintenir deux obligations phares de la loi Égalité et citoyenneté que vous avez supprimées

soutient le souhait du Gouvernement de ne pas modifier l'équilibre actuel de la loi SRU. M. le ministre l'a rappelé, cette loi de 2000 est un outil de mixité sociale qui fonctionne bien au regard des quelque 250 communes carencées. Certains problèmes demeurent à la marge, mais sont généralement réglés par les préfets. Il importe de garder ce cadre général pour construire du logement social. C'est pourquoi nous nous opposerons aux mesures d'assouplissement et d'expérimentation adoptées en commission. Mes chers collègues, ne soyons pas dogmatiques, ne faisons pas la loi au travers d'exemples personnels : l'enjeu est trop important pour nos concitoyens. La parole

la question du logement est aujourd'hui fondatrice et structurante : il s'agit de savoir dans quelle société nous voulons vivre. Avoir un toit, est-ce encore un droit ? Telle est la question, quand on voit que vous considérez le logement comme un produit marchand, source de spéculation, de placements et de stratégies financières. L'habitat, ce n'est pas simplement un produit pour promoteur ou une source de revenus pour ceux qui ont investi dans la pierre. De la qualité du logement, de sa taille, de sa configuration dans son environnement, de sa proximité avec les services publics en fonction de la mixité de l'espace dépendra, pour beaucoup, la qualité de vie de ses occupants.

Ainsi, le logement et sa qualité ont un rôle fondamental pour l'aménagement du territoire de notre pays. Au-delà, parce qu'il a une incidence considérable sur l'épanouissement de chacune et de chacun, l'habitat joue un rôle fondamental dans le vivre en société, dans le faire ensemble.

celle d'un nouveau monde qui confond intérêt général et ambition pour l'avenir avec une gestion à la petite semaine en mode start-up branchouille ; celle d'un Gouvernement qui confond les coups de com'à répétition avec l'exigence d'agir pour les décennies à venir. Le projet de loi, dans la foulée de la loi de finances pour 2018, n'a qu'un prisme : réduire l'engagement public du secteur du logement. Avec ce énième désengagement, un pactole est en perspective pour les lobbies de l'immobilier, qui gagnent ici le droit de construire plus vite, moins bien et souvent plus cher

Par ce projet de loi, le Gouvernement mène une attaque en règle contre le modèle même du logement social. En effet, le logement social, dans notre pays, repose sur trois piliers : il s'agit d'un bien public, qui fait l'objet d'une cogestion avec les habitants, au plus près du territoire, par l'intermédiaire d'organismes d'HLM à taille humaine pilotés par les élus de ce territoire. D'un revers de main, vous revenez sur tous ces fondements. Vous obligez à la vente en masse, y compris dans les communes carencées au titre de la loi SRU, vous obligez au regroupement des offices et vous évincez les représentants des locataires de ces nouvelles structures.

offices doivent également composer avec la quasi-suppression des aides à la pierre. Comment, demain, pourront-ils produire l'effort nécessaire pour répondre à la demande ? Soyons clairs : la vente de logements sociaux aujourd'hui, c'est l'explosion du mal-logement demain. Ce sont des copropriétés dégradées et le patrimoine récent vendu au privé pour un plus grand retour sur investissement, notamment dans les zones les plus demandées. Or, jusqu'ici, personne n'avait osé soustraire ce patrimoine

Après avoir flexibilisé le droit du travail, vous flexibilisez le bail, par le bail mobilité. Toute volonté de régulation a été supprimée, notamment l'encadrement des loyers, ou encore la garantie universelle des loyers, qui s'est transformée en garantie spécifique VISALE. Or tous les indicateurs sont au rouge. Le poids des dépenses de logement dans le budget des ménages continue de peser trop lourd, et la rente immobilière ne faiblit pas, avec des niveaux de loyers toujours trop élevés. Pourtant- « en même temps », devrait-on dire -, ce gouvernement n'en finit plus d'économiser sur les aides au logement. plus utile pour financer les crédits d'impôt et autres niches fiscales sans même les évaluer, afin de conserver celles qui ont un effet levier et de supprimer les autres. Votre seul choix, c'est de retirer au logement public pour financer l'investissement privé sans souci des conséquences territoriales. Bien sûr, nous regrettons que le passage en commission ait encore aggravé ce texte par une remise en cause inacceptable de la loi SRU, mettant au ban la nécessaire solidarité territoriale. loi, on ne trouve rien sur les quartiers, malgré les propositions du plan Borloo ; rien sur les territoires ruraux et l'effort gigantesque à produire en termes de réhabilitation ; rien non plus sur les zones dites « détendues » ; rien sur l'impérieuse obligation qui est la nôtre d'apporter des solutions pour éviter des désertifications territoriales et une dégradation de l'existant ; rien sur la réimplantation de circuits courts de production de matières premières pour la construction, permettant de penser l'habitat de demain, de relever les défis environnementaux du secteur du bâtiment et de créer des emplois non délocalisables. Alors, je le réaffirme ici fortement, nous considérons que nous avons plus que jamais besoin d'une politique publique du logement pour répondre aux besoins de nos concitoyens, des plus jeunes aux plus âgés. Ils sont près de 2 millions à attendre un logement social, près de 12 millions à souffrir d'une manière ou d'une autre du mal-logement. Pour eux, il n'y a aucun gâteau à partager : toutes les parts iront aux plus aisés, aux plus chanceux. Par nos amendements, nous tenterons d'apporter des solutions et des pistes pour une politique du logement progressiste, humaniste, à l'inverse de votre logique de financiarisation et de privatisation de ce bien de première nécessité, de cet élément consubstantiel de la dignité qu'est le fait d'avoir un toit.

C'est au terme d'un long processus que nous abordons aujourd'hui l'examen du projet de loi ÉLAN. Je salue à ce titre l'implication du Sénat et de son président, Gérard Larcher, à l'initiative de la conférence de consensus, qui a permis de recueillir, auprès des professionnels du logement et de l'aménagement, un nombre de propositions digne de l'ampleur du texte proposé par le Gouvernement. Au travers des interrogations soulevées par les acteurs rencontrés lors de cette conférence comme au cours du travail préparatoire qui a suivi, de grands enjeux ont pu être identifiés, qui conditionnent l'examen du projet de loi. Tout d'abord, la place des collectivités est rapidement apparue comme une problématique centrale. Celle-ci est en effet remise en cause tout au long du texte, et ce au profit d'une recentralisation, à rebours du discours de prise en main des politiques locales par les acteurs locaux, pourtant attendue et soutenue. La gouvernance territoriale est essentielle. Nous défendrons des propositions en ce sens, pour que les politiques du logement et de l'habitat soient opérationnelles à une échelle pertinente sur le territoire et adaptées aux réalités locales. Sans surprise, l'impact de la loi de finances pour 2018 et de la réduction de loyer de solidarité ne peut être occulté. Cette mesure a d'ores et déjà profondément affecté l'activité des bailleurs sociaux et le nombre de logements produits. Or le projet de loi ÉLAN ne nous semble pas permettre de remédier à l'ensemble des difficultés constatées.

pour atteindre les objectifs de l'article 55 de la loi SRU, dont nous ne voulons pas le détricotage, mais pour lequel le principe de réalité doit s'appliquer, car des distorsions et des phénomènes contradictoires se nous vous rejoignons dans la volonté de réformer le secteur du logement social. Vos objectifs sont louables, et nous les approuvons. Toutefois, les moyens que vous comptez mettre en oeuvre pour les atteindre ne nous paraissent, souvent, adaptés ni aux besoins des bailleurs ni aux intérêts des habitants de ces logements. Vous proposez ainsi de regrouper les organismes de logement social afin de gagner en efficacité de gestion et de dégager des économies. Or vous risquez parfois de créer des structures surdimensionnées, sans prise avec les réalités fines de nos territoires, même si, comme vous l'avez rappelé,

Vous proposez également de remédier à la baisse des aides publiques au logement en faisant de la vente du parc social un moyen de financement. Vous ouvrez ainsi la voie à une privatisation dangereuse du secteur. Vous fixez même un objectif annuel de vente de 40 000 logements sociaux par an, alors même que- vous l'avez rappelé -l'ensemble des bailleurs réunis ne dépassent cette vente ne peut être menée dans une seule logique comptable, sans accompagnement des reprises de logements. Nous devons anticiper la constitution de copropriétés dégradées et être particulièrement vigilants

se voient remettre, à l'échelle territoriale, la mise en oeuvre des politiques voulues par le Gouvernement. Outre les dangers qu'elles impliquent pour l'avenir de l'ensemble du secteur, ces mesures s'ajoutent à d'autres évolutions récentes qui consacrent le retour de l'État central et où l'idée de coproduire les politiques publiques avec les acteurs territoriaux disparaît, qu'il s'agisse des politiques de l'habitat ou de l'aménagement du territoire. À ce titre, la réforme d'Action logement est particulièrement révélatrice. Les mesures proposées relèvent d'une même logique, d'une même philosophie, que nous ne saurions approuver sans que certains engagements de l'État soient réintroduits.

du secteur du logement, des associations de locataires et des élus. Ladite conférence a permis à tous les participants de s'exprimer, dans le respect de chacun, et d'identifier des lignes de convergence. le rôle des élus dans la politique du logement, la simplification du droit de l'urbanisme et des normes de construction, la nécessaire mobilisation du foncier, la revitalisation des centres-villes sont autant de sujets qui font consensus, ici, au Sénat. Le groupe socialiste avait alors affirmé ses orientations autour de trois préoccupations majeures : la nécessité d'une politique du logement au plus près des des territoires, la modernisation sans altération du modèle du logement social et la qualité de vie pour tous nos concitoyens. Permettez-moi d'associer à ce propos notre collègue Annie Guillemot, qui ne peut malheureusement pas être avec nous cette semaine pour des raisons de santé, mais qui a accompli un important travail sur ce texte, lors des auditions, à nos côtés. Le projet de loi, notamment son titre I, sur lequel je concentrerai mon propos, affiche des objectifs que nous aurions pu soutenir sans aucune difficulté, tel que « construire plus, mieux et moins cher quelques désaccords quant aux moyens nous en empêchent. Le projet de loi propose aux collectivités de nouveaux outils de contractualisation, les PPA ou encore les GOU, pour engager des opérations d'aménagement complexes en associant tous les partenaires publics et privés. Au-delà de la nécessaire prudence qu'il convient d'observer quand on légifère à nouveau, singulièrement dans le domaine de la construction et de l'aménagement,

dans la proposition de loi que nous avions présentée et que le Sénat avait adoptée à l'unanimité. Mais le projet de loi issu de l'Assemblée nationale comporte des mesures qui contraignent et dessaisissent le maire d'une compétence majeure. Nous y sommes résolument, définitivement opposés. nous aurons ce débat à propos de vos amendements. Notre conviction est qu'il faut agir dans la coconstruction et non dans la confiscation. Le transfert de la compétence « permis de construire », par exemple, est une disposition qui est contraire à l'intérêt des territoires et à l'efficacité d'une bonne mise en oeuvre des politiques publiques. De plus, ce qui pourrait s'apparenter à une méfiance envers les élus locaux, à un manque de confiance

En effet, depuis l'automne, les bailleurs sociaux ont fait leurs comptes : les mesures de contrepartie à la baisse des loyers adoptées en loi de finances ne compenseront pas, loin de là, la chute de leur autofinancement.

Construire plus, mieux et moins cher, mais avec moins de moyens : voilà donc le pari risqué du Gouvernement. Nous allons essayer pendant cette longue semaine, à travers de multiples dispositions, de redonner un peu d'oxygène au secteur, mais sans moyens budgétaires. Vous comptez d'abord sur la réorganisation des bailleurs sociaux, dont vous attendez des économies d'échelle. C'est évidemment possible, mais à quelle hauteur ? Toute la question est là. Quant à la vente de logements sociaux, autre mesure phare de votre réforme, l'objectif de 40 000 logements par an me semble inatteignable, malgré les montages financiers que vous imaginez, sans parler de ceux dont rêvent certains, mais qui conduiraient à une quasi-privatisation d'une partie du secteur du logement social, dont j'espère bien que nous tuerons dans l'oeuf, ici, au Sénat, toute velléité. la disposition issue de ce que certains ont appelé l'« amendement Monopoly », relatif à l'usufruit locatif social, étonnamment adopté sans aucun débat à l'Assemblée nationale et avec un surprenant avis favorable du Gouvernement.

en prenant les précautions nécessaires pour protéger les locataires et les futurs acquéreurs, il serait inacceptable que cela se fasse au bénéfice d'intérêts privés profitant d'un bel effet d'aubaine : l'assèchement des finances des bailleurs, organisé par l'État lui-même. Le capital que représentent ces logements, financés en grande partie sur fonds publics, s'il peut être mobilisé, doit évidemment rester dans le giron public. public. Au-delà des aspects financiers, il faut également bien mesurer le risque que la vente d'HLM représente, car, à l'évidence, les logements que l'on vendra seront les mieux situés, les mieux entretenus et ceux dont les locataires en auront les moyens. Concentrer à nouveau les ménages les plus pauvres ou en prendre le risque serait une grave erreur en matière de mixité sociale, bien sûr, mais également pour l'équilibre des budgets des bailleurs. Espérons donc qu'ils manieront cet outil avec précaution et surtout que nos communes, en particulier les maires, seront étroitement associées aux prises de décisions, pour en limiter les conséquences. Quant à la circulation des capitaux au sein des nouvelles entités, sociétés anonymes de coordination ou groupes, elle sera certes utile, mais ce n'est pas parce que nous aurons branché de nouveaux tuyaux que la source des financements que vous aurez contribué à réduire retrouvera son débit précédent Voilà pourquoi je suis persuadé qu'il ne sera pas possible de construire plus. Je doute même que nous soyons en mesure de construire demain autant qu'au cours des deux dernières années. le ministre, monsieur le secrétaire d'État, pour ajuster votre ambition à la situation que vous allez créer, de la limiter à cette formule : construire au moins autant, mieux et moins cher, avec moins de moyens. Si nous y parvenions, ce serait déjà un beau résultat. Comment, en effet, ne pas s'inquiéter du nombre de logements sociaux financés en 2017 ? À 113 000, il a déjà marqué une inflexion par rapport aux 126 000 de 2016. Chacun sait que c'est au dernier trimestre que le chiffre de l'année se construit, lorsque les dossiers sont remontés du terrain et que l'ajustement de la répartition des aides à la pierre est opéré par le FNAP. Au reste, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État,

Pendant ce temps, les maires, qui portent les objectifs de construction que l'État leur assigne, par exemple au travers de l'article 55 de la loi SRU, ou ceux inscrits dans les schémas régionaux ou intercommunaux, vont se retrouver entre le marteau et l'enclume. Vente d'HLM d'un côté, opérateurs disposant de moins de moyens de l'autre, collectivités territoriales aux budgets fortement contraints il ne faudra pas oublier, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, la part de responsabilité qui aura été la vôtre, si jamais les objectifs ne sont pas atteints. Certes, notre pays doit réaliser des économies pour revenir à l'équilibre budgétaire et inverser enfin la courbe de la dette publique. Mais, pour ce faire, fallait-il s'attaquer ainsi, avec une telle brutalité, à ce secteur d'activité ? Je ne le crois pas. Oui, la France consacre plus de 40 milliards d'euros par an à la politique du logement, dont près de la moitié est destinée aux aides personnelles, qui sont, je le rappelle, les aides les plus redistributives de notre système social Le Président de la République a appelé, lors du dernier Congrès à Versailles, à la construction de « l'État providence du XXI siècle ». Belle formule ... Mais que recouvrera-t-elle vraiment ? En ce sens, le secteur du logement aurait dû rester une priorité. Il ne l'est plus, sauf pour Bercy, mais qui n'y voit que l'un des premiers postes d'économies possibles. Pourtant, aussi bien pour la croissance et les rentrées fiscales qu'il engendre que pour l'emploi non délocalisable qu'il procure, le secteur du logement est essentiel au dynamisme de notre économie. Pour les Français, le logement est, comme l'emploi, une préoccupation centrale. De fait, un logement digne et abordable est l'une des conditions essentielles de la construction d'un projet de vie, l'une des conditions essentielles de la réussite scolaire des enfants des familles les plus modestes, l'une des conditions essentielles de la cohésion sociale.

réduire le montant des aides personnelles, comme vous vous apprêtez à le faire de nouveau, pour près de 1 milliard d'euros, si j'ai bien compris, dans la prochaine loi de finances, serait prendre le risque d'aggraver les difficultés des ménages les plus pauvres. C'est vrai ! L'autre moitié de ces 40 milliards est consacrée, directement ou indirectement, aux aides à la construction. Les réduire, c'est prendre le risque de voir chuter le nombre de logements construits, y compris en accession à la propriété, car, aujourd'hui, de nombreuses opérations sont mixtes c'est pénaliser la classe moyenne, qui est déjà la grande oubliée de votre politique depuis le début de ce quinquennat. Un mot, pour terminer, de l'article 55 de la loi SRU. Tout le monde sait- en tout cas ceux qui ont un jour exercé des responsabilités locales -que l'objectif de 25 % de logements sociaux en 2025 est inatteignable pour nombre de communes, même pour celles qui ont jusqu'ici parfaitement respecté la loi et n'ont donc jamais été carencées.

le CGEDD préconise le recrutement de fonctionnaires dans les préfectures ... Ah non ! ... pour gérer, en lieu et place des maires, le droit de préemption des communes et la mise en oeuvre de toutes les sanctions prévues par la loi- vous savez qu'elles sont nombreuses. Cela, mes chers collègues,

des accommodements raisonnables qui, sans dénaturer l'esprit de la loi, permettraient de l'adapter aux diverses situations de nos territoires ? Il le faut, car rien ne serait pire que de décourager définitivement les maires qui sont engagés dans la construction de logements sociaux, contrairement à la poignée de ceux qui ne veulent rien faire et le proclament haut et fort.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'encouragement à concentrer les activités économiques dynamiques dans les métropoles a contribué, comme notre groupe l'a toujours souligné lors des réformes territoriales, à accentuer les fractures territoriales et, incidemment, la crise du logement. Cette situation illustre malheureusement l'accroissement des inégalités dans les villes et leur périphérie, comme dans la ruralité. De façon générale, nos concitoyens aspirent à juste titre à un meilleur cadre de vie, mais également à un accès équitable aux services publics, aux transports et aux activités culturelles, quel que soit leur lieu d'habitation. Certes, quelques évolutions changent petit à petit la donne : nouvelles mobilités, télétravail, développement de l'autoentrepreneuriat, organisation par les entreprises des déplacements de leurs salariés. Autant de tendances qui réduisent les tensions sur le logement dans les grandes agglomérations. Pour autant, la succession des lois a surtout donné l'impression d'une cohésion territoriale inatteignable. Le présent projet de loi apporte, à notre sens, des réponses pragmatiques et concrètes, qui correspondent aux attentes. J'en évoquerai quelques-unes dans le temps qui m'est imparti. L'accès au logement passe incontestablement par un renforcement de l'offre, alors que les normes de construction ont connu une inflation de 60 % au cours de la dernière décennie. La volonté de simplifier est indispensable, afin de donner une lisibilité aux normes et de faciliter l'innovation par la numérisation. Dans le même esprit, nous soutiendrons des mesures fortes et attendues libération du foncier public, transformation des bureaux vacants en logements, création de grandes opérations d'urbanisme, dématérialisation de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et lutte contre les recours abusifs. Nous approuvons également les dispositions qui renforcent le rôle du parc social, tout en encourageant la rotation, notamment en Île-de-France. Dans son rapport public la Cour des comptes a signalé que 48 % des ménages résidant dans les logements sociaux ne sont ni modestes ni défavorisés, ce qui tend à évincer le public prioritaire. Or cette situation concerne la moitié des ménages situés sous le seuil de pauvreté. L'accès au logement social doit donc avoir lieu dans des conditions justes et mieux adaptées aux capacités financières des locataires. Le projet de loi va dans ce sens, en généralisant la cotation de la demande pour accroître la transparence des attributions. Enfin, monsieur le ministre, je vous sais soucieux d'élargir l'accès à la propriété des Français, dans un contexte de mobilités accrues et de nouvelles formes de travail. Plus globalement, le projet de loi est l'occasion d'apporter à nos concitoyens de nouvelles garanties sur un sujet au coeur de leurs préoccupations quotidiennes. Vous l'aurez compris, notre groupe porte un regard très favorable sur ce texte, qui ne crée pas de contraintes supplémentaires et rejoint les principes que nous défendons depuis des années, dans un souci de pragmatisme et de simplification. Nous veillerons donc scrupuleusement à ce qu'il ne soit pas dénaturé. La parole

nous voici réunis pour examiner le projet de loi dit ÉLAN, qui porte sur un sujet crucial pour notre société : la crise du logement.

Dominique Estrosi Sassone, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Leleux et Patrick Chaize, pour le travail qu'ils ont accompli. Leur tâche n'était pas facile, compte tenu du peu de temps qui nous a été accordé pour travailler sur ce projet de loi. Monsieur le ministre, le 14 juin dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité des suffrages exprimés, par 288 voix pour et aucune contre, la proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,

Quoi qu'il en soit, l'adoption unanime de ce texte est la preuve qu'il fallait s'attaquer aux fléaux qui rongent nos coeurs de ville. Nous le faisons ! Je ne reviendrai pas sur son contenu. Toutefois, avec notre collègue Martial Bourquin, coauteur de la proposition de loi, je me réjouis que la commission des affaires économiques ait inscrit dans son texte les dispositions que nous jugeons nécessaires pour mettre un terme à la culture de la périphérie

de réduire le seuil d'autorisation d'implantation commerciale, cette fois dans les périmètres ORT, et non OSER. Vous voyez, monsieur le ministre, que nous sommes conciliants aussi un processus de délivrance d'installation commerciale soumis à une étude d'impact, qui devra tenir compte du tissu économique existant. En somme, ces mesures forment un ensemble cohérent, avec des objectifs fixés par le pacte national, au service de la reconquête de nos centres-villes au sens large- car l'enjeu n'est pas seulement commercial, mais également urbanistique. Il faut que les habitants se réapproprient les coeurs de ville, pour que ceux-ci se repeuplent. Nous étions également dépositaires de plusieurs amendements examinés en commission. Nous avons choisi de ne proposer que des dispositions susceptibles d'être conjuguées avec celles que vous nous proposez, conformément à l'esprit de la conférence de consensus sur le logement voulue par le président du Sénat, Gérard Larcher. Ainsi, nos dispositions visant à rééquilibrer la fiscalité entre commerces de proximité, de périphérie et électronique n'ont pas fait l'objet de nouveaux amendements, à l'exception d'une mesure, qui donnera lieu à un amendement d'appel destiné à rappeler que, sans de nouvelles recettes fiscales, nous ne pourrons absolument rien faire. Je connais les réticences de Bercy et des commissions des finances.

le secrétaire d'État, mes chers collègues, le Sénat est mobilisé pour faire bouger les choses. Contrairement à certaines idées reçues, nous sommes des progressistes, mais des progressistes soucieux d'aller dans le bon sens. C'est dans cet esprit que nous vous présenterons d'autres amendements.

petites villes de France -, mais également par les associations professionnelles de commerçants. Ne les décevons pas ! Donnons des raisons d'espérer à nos millions de compatriotes qui vivent dans des villes et villages trop souvent délaissés et conservons la place des collectivités territoriales,

où et comment générer la ville à travers la construction de logements ? Pour qui construit-on ? Comment répartir la population sur un territoire en tenant compte des mobilités et des infrastructures ? Comment protéger la qualité de vie en construisant du logement de qualité ? On voit bien là le rôle primordial des collectivités territoriales et des élus locaux. C'est sur eux que s'appuient les politiques de l'habitat. Le projet de loi ÉLAN vise à construire plus, mieux et moins cher. Son objectif apparaît essentiellement quantitatif. Mais un logement, c'est avant tout un lieu de vie intime : on s'y sent bien à condition qu'il corresponde à ses aspirations et que l'environnement vu depuis sa fenêtre, ou lorsque l'on sort de chez soi, est source de bien-être. Voilà pourquoi les architectes et les architectes des Bâtiments de France, en liaison avec les urbanistes et les paysagistes, ont un rôle majeur à jouer en matière de construction de logements. C'est pour cela que la commission de la culture du Sénat et son rapporteur pour avis, Jean-Pierre Leleux, se sont attachés à remettre la dimension qualitative au coeur du projet de loi. En effet, construire vite et moins cher ne saurait se substituer à construire bien le paysage, qu'il soit urbain ou non. Le patrimoine, les espaces verts et publics, la qualité architecturale sont autant d'éléments nécessaires à la qualité de vie à laquelle tous nos concitoyens aspirent. Ils doivent donc être au coeur du projet.

Veiller aux commerces, aux services et à la qualité de vie est une condition essentielle pour redonner envie de vivre dans le coeur de nos villes et de nos bourgs ! Nous soutiendrons donc cette vision globale, clé d'une politique du logement réussie. Toutefois, de grands défis se présentent encore à nous : le mal-logement, la précarité croissante, la dégradation du parc ancien à réhabiliter, la lutte contre l'étalement urbain, la désertification rurale, le vieillissement, les nouveaux besoins des familles, le retour de la nature en ville, le retour de la mixité sociale dans de nombreux quartiers, et j'en passe. Ces défis, il va bien falloir y répondre de manière globale, coordonnée et avec un financement. Ce sera forcément sur le terrain, avec les collectivités territoriales, les élus locaux, les acteurs de la construction et les habitants que cela se jouera.

pour une meilleure adéquation entre les besoins quantitatifs et qualitatifs des citoyens et ceux des territoires et des collectivités territoriales. Bien construire du logement, c'est bien construire notre société et permettre à chacun de bien se construire.

monsieur le ministre, votre stratégie pour le logement, j'ai pu constater des ambitions et des objectifs que nous avions en partage : la relance de la construction pour répondre aux besoins de logement, la rénovation urbaine pour améliorer le cadre de vie, la volonté de favoriser l'accession à la propriété dans le cadre d'un parcours résidentiel efficace.

la trahison des actes sur les mots a débuté bien avant ce projet de loi ; elle s'est révélée, voilà quelques mois, dès la présentation du projet de loi de finances pour 2018 et des moyens budgétaires pour le logement diminution des aides à la pierre, diminution des APL, suppression de l'aide aux maires bâtisseurs, déstabilisation majeure du modèle du logement social par la suppression de 70 % de la capacité d'investissement des organismes d'HLM ... Dans un pays où plus de 4 millions de personnes souffrent du mal-logement, il est inacceptable de freiner la construction de logements ! Inacceptable de demander aux plus modestes de se serrer la ceinture, quand les plus aisés bénéficient des largesses fiscales du pouvoir

Aujourd'hui, le projet de loi que nous examinons est vicié par l'idée centrale sur laquelle il repose : celle qui consiste à considérer la politique du logement comme une politique coûteuse pour la Nation. Partir de ce constat, c'est oublier sciemment les ressources qu'elle apporte en termes de TVA, de taxe foncière et d'activité économique. Investir dans le logement, c'est investir pour que chacun ait un toit ; c'est investir dans le secteur du bâtiment, le premier employeur de France. C'est donc ferrés par le dogmatisme de Bercy que nous allons débattre, alors que nous aurions pu construire ensemble des solutions de logement réconciliant humanité, solidarité et économie. Le projet qui nous est présenté s'inscrit dans une logique de centralisme, de privatisation et de financiarisation du patrimoine français du logement social, au détriment de la mixité sociale et de l'accès au logement pour tous. En limitant la capacité financière des bailleurs HLM et en les regroupant, monsieur le ministre, vous les contraignez à s'orienter vers le secteur privé pour emprunter. Vous autorisez la vente en bloc d'immeubles HLM, alors que vous avez avoué, la semaine dernière, que les objectifs en termes de construction de logements sociaux seront difficiles à atteindre. Croire que vendre une HLM permettrait d'en construire trois est bel et bien un fantasme : l'expérience a toujours montré que la vente de logements HLM ne se substitue pas à l'investissement de fonds publics pour construire davantage de logements sociaux. Aborder la thématique du logement, c'est prendre à bras-le-corps la question de la mixité sociale et le devoir républicain de garantir à tous la possibilité d'être logé. En commission, la majorité sénatoriale l'a oublié. En dévitalisant avec méthode la loi SRU, elle a profondément attaqué cette mixité, en dépit de toute logique de justice et de bon sens économique. Comptabilisation dans les 25 % de logements sociaux des logements provisoires, passage de 1 500 à 3 500 habitants pour l'exemption des communes en Île-de-France

Concentrer la pauvreté dans certaines villes et dédouaner certaines autres de leur devoir de mixité sociale, voilà votre projet ! Qu'il s'agisse des 100 % de logements accessibles ou du respect de la loi SRU, vous pensez vous attaquer à des dogmes de la gauche ; mais c'est avant tout à des nécessités de notre République Contrairement à ce que vous laissez penser, ces règles ne sont pas maximalistes. Des dérogations sont prévues, qui prennent en compte les réalités du terrain. Ainsi, plus de la moitié des communes françaises sont exemptées de la loi SRU, et, parmi celles qui ne respectent pas leurs obligations, 250 seulement sont déclarées carencées. Le

l'accessibilité ne peut pas être réduite à des considérations techniques. Je comprends la volonté de Mme la rapporteur de trouver un compromis avec le Gouvernement, mais l'accessibilité ne peut pas faire l'objet de solutions de compromis, car elle conditionne la concrétisation des droits des personnes handicapées, mais aussi dépendantes ; elle est un préalable nécessaire à leur participation sociale. C'est pourquoi nous défendrons avec force le maintien de l'obligation de 100 % de logements accessibles.

c'est tout faire pour éviter de foncer tête baissée dans l'impasse d'une durable cohabitation entre « ghettos de riches » et « ghettos de pauvres ». Mes chers collègues,

pas à la réalité. Je vais en donner quelques exemples. En quoi ce texte met-il en danger le pouvoir exécutif des maires ?

Que trouve-t-on dans ce texte ? La création des PPA et des grandes opérations d'urbanisme, qui ne visent que des dossiers lourds d'aménagement d'aménagement voulus par les collectivités locales. C'est pour faciliter le travail des collectivités locales qui le demanderont que nous avons mis en place

ont donc un impact. Surtout, ces dispositifs sont entièrement confiés à la responsabilité des maires, à tel point, d'ailleurs, que le comité de projet mis en place dans chaque territoire retenu est présidé

du pouvoir des maires et des collectivités locales

Mes chers collègues, par lettres en date des 12 et 13 juillet 2018, M. Patrick Kanner, président du groupe socialiste et républicain, et Mme Éliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ont demandé que le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière soit examiné selon la procédure normale et non selon la procédure simplifiée. En conséquence, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande que ce projet de loi, dont l'examen était initialement prévu le jeudi 19 juillet, soit inscrit à l'ordre du jour du jeudi 26 juillet, à dix heures trente. Acte est donné de ces demandes. Dans la discussion générale, le temps attribué aux orateurs des groupes sera d'une heure. Le délai limite pour les inscriptions de parole est fixé au mercredi 25 juillet, à quinze heures. Il n'y a pas d'opposition ? ... Il en est ainsi décidé. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein d'une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges.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

Monsieur le président, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis de l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi, qui vise à interdire l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges. Vous le savez, ce texte concrétise un engagement de campagne du Président de la République. Je suis évidemment fier, en tant que ministre de l'éducation nationale, de pouvoir mettre en oeuvre L'interdiction du téléphone portable répond à des enjeux à la fois éducatifs et de vie scolaire. Durant les activités d'enseignement, l'interdiction de l'usage des téléphones portables permettra de garantir aux élèves un environnement propice à l'attention, à la concentration, à la réflexion, indispensable à l'activité, à la compréhension et à la mémorisation. Sur les temps de récréation, l'usage du téléphone portable peut s'avérer néfaste en réduisant l'activité physique et en limitant les interactions sociales entre les élèves- nous pouvons déjà en faire le constat en comparant les collèges qui ont décidé d'instaurer une telle interdiction et ceux qui ne le font pas. Cet usage peut empêcher la construction d'une sociabilité harmonieuse, essentielle au développement des enfants. Les chefs d'établissement le disent unanimement : une cour sans téléphone portable, c'est une cour où les enfants jouent, discutent, chahutent, où ils vivent leur vie d'enfant. Par ailleurs, l'usage des téléphones portables est à l'origine d'une part importante des incivilités et des perturbations dans les établissements : casses, rackets, vols. Ils servent aussi souvent de supports aux phénomènes de cyberharcèlement, lesquels exportent la violence, de surcroît, en dehors des établissements. Les téléphones portables peuvent en outre faciliter l'accès aux images violentes et aux images pornographiques. L'interdiction de l'usage du téléphone portable constitue l'un des outils susceptibles de limiter l'exposition des plus jeunes à des images choquantes.

Ce constat me semble aujourd'hui partagé par tous ; certains d'entre vous s'interrogent toutefois sur la nécessité de légiférer, au motif que l'interdiction du téléphone portable à l'école est d'ores et déjà en partie dans le code de l'éducation. Je souhaite répondre à cette interrogation, qui me paraît légitime. En l'état actuel du droit, l'article L. 511-5 du code de l'éducation prévoit l'interdiction de l'usage des téléphones portables durant les heures d'enseignement et dans les lieux qui sont prévus par le règlement intérieur. Cependant, le juge administratif n'admettant pas de manière certaine la légalité d'une interdiction générale prise par le pouvoir réglementaire, et seuls les chefs d'établissement pouvant inscrire à l'ordre du jour des conseils d'administration une telle mesure sans que cela soit considéré comme un impératif, l'effectivité de cette interdiction n'est aujourd'hui pas assurée. C'est donc bien la volonté de garantir l'interdiction effective de l'utilisation du téléphone portable dans toutes les écoles et dans tous les collèges qui justifie cette proposition de loi. Je souhaite loi. Je souhaite également saluer la souplesse que permet ce texte quant à la mise en oeuvre pratique de l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables. J'y suis évidemment très sensible, en tant que ministre de l'éducation nationale. La rédaction actuelle de l'article 1 donne la possibilité au règlement intérieur de chaque établissement de préciser les modalités de cette interdiction. Contrairement à ce qu'il m'est arrivé d'entendre, il n'est pas question d'imposer des casiers dans tous les établissements, mais, tout simplement, de permettre qu'une telle Chaque établissement, en fonction de la configuration de ses locaux et de son organisation propre, pourra définir les modalités d'application de cette interdiction, au plus près de ses spécificités. Le ministère publiera prochainement, dès que la proposition de loi sera adoptée, un vade-mecum élaboré par les services de la DGESCO, avec l'appui d'un groupe de travail réunissant notamment des professeurs et des chefs d'établissement, tenant compte de nos débats, pour accompagner les établissements dans la mise en oeuvre concrète de cette interdiction. Ce document présentera également les bonnes pratiques. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement, que je représente aujourd'hui, accueille très favorablement cette proposition de loi, que je vous invite donc à adopter très largement. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne vous cacherai pas que, lorsque j'ai été nommé rapporteur de cette proposition de loi par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, mes premières réflexions furent pour m'interroger sur le bien-fondé de ce texte.

L'application d'un programme électoral, fût-il présidentiel, ne me pose aucun problème. Encore faut-il que cette application corresponde à un vrai besoin, particulièrement en ces temps où l'on nous propose de réviser la Constitution, avec pour objectif, notamment, de légiférer mieux et moins. La perception par l'opinion publique est plus nuancée qu'il n'y paraît au premier abord, et, monsieur le ministre, il ne faudrait pas interpréter l'enthousiasme général que chacun d'entre nous a pu observer, ces dernières heures, dans les rues de tout le pays comme une adhésion profonde à cette initiative. Certes, les parents et les enseignants l'accueillent plutôt avec bienveillance, mais ils ne manquent pas de faire observer qu'il est plus facile d'interdire le téléphone portable dans les écoles et les collèges que dans les prisons, où leur utilisation constitue pourtant un vrai problème. Si beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, estiment que les dispositions de cette proposition de loi ne relèvent pas du domaine de la loi, c'est parce qu'il existe déjà des dispositions législatives à ce sujet, et que ces dispositions sont perfectibles. Introduit par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, d'ailleurs sur l'initiative du Sénat, l'article L. 511-5 du code de l'éducation interdit l'utilisation par un élève du téléphone portable « durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur La loi de 2010 obéissait donc à une autre logique, celle de la protection des élèves des ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, nous sommes amenés, en quelque sorte, à revoir notre copie, mais dans une tout autre perspective, celle de la vie scolaire et de la réussite des élèves.

D'abord, leur utilisation perturbe les enseignements et constitue un facteur d'indiscipline en classe. La sollicitation permanente des élèves a des conséquences directes sur leurs capacités d'attention et d'apprentissage : aucun élève ne peut en même temps prêter pleinement attention au professeur au professeur et envoyer des messages sur son smartphone ! Ensuite, il faut évoquer les conséquences parfois graves de l'utilisation de ces appareils : prises de vue sans consentement, harcèlement sur internet, exposition à la pornographie. Du fait de leur prix, ils sont en outre l'objet de vols et de querelles. Enfin, alors que l'école est un lieu de sociabilité, l'usage du smartphone alimente le repli sur soi de certains élèves. Les auditions que j'ai menées permettent de conclure que, lorsque l'utilisation des téléphones portables a été interdite dans toute l'enceinte de l'établissement, comme c'est déjà le cas dans certains endroits, cela s'est traduit par des conséquences positives tant sur les apprentissages que sur le climat et la vie scolaires. La simplicité et la lisibilité de l'interdiction facilitent son appropriation par les élèves et leurs parents ; son extension à l'ensemble de l'établissement s'est traduite par un moindre nombre d'incidents en classe, où l'usage était déjà interdit, et par un moindre nombre de confiscations. En outre, le climat scolaire s'est amélioré, et l'on observe une plus grande socialisation entre élèves, les jeux de ballon faisant par exemple leur retour dans les cours d'école. Pour en revenir au cadre juridique, l'article L. 511-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur, présente deux défauts majeurs. Premièrement, parce qu'elle distingue les activités d'enseignement, pendant lesquelles l'utilisation du téléphone portable est interdite, des autres temps de présence dans les établissements, cette disposition ne permet pas au règlement intérieur d'interdire l'utilisation du téléphone portable de manière générale et absolue ; hors de la classe, la liberté d'usage doit demeurer la règle. Si un grand nombre d'écoles et de collèges, dans des proportions que le ministère est incapable de mesurer, mettent en oeuvre cette interdiction, la légalité de cette mesure est très fragile et, dans certaines académies, les services juridiques des rectorats s'y opposent. Deuxièmement, parce qu'il interdit de manière absolue toute utilisation du téléphone portable pendant les activités d'enseignement, l'article L. 511-5 place les établissements et les enseignants ayant recours

Cela est problématique, dans la mesure où le BYOD tend à se développer. Un certain nombre de collectivités territoriales envisagent en effet d'y recourir, afin de rompre avec les politiques d'équipement de l'ensemble des élèves, très coûteuses et souvent peu efficientes. Se pose également la question de la confiscation, qui constitue, après la réprimande, la solution la plus courante pour mettre fin à une utilisation illicite du téléphone portable. Son cadre juridique est incertain et fait l'objet d'interprétations contradictoires. Si elle est largement pratiquée, elle n'est mentionnée dans les circulaires ministérielles que dans le cas d'objets dangereux ou toxiques, ce que ne sont évidemment pas les téléphones portables. Notons qu'il est écrit, sur le site service-public.fr, que « la confiscation du téléphone portable n'est pas autorisée Les chefs d'établissement et les enseignants rencontrés nous ont fait part de leur souhait de voir sécurisées leurs pratiques et clarifié ce cadre juridique, d'autant que la confiscation est souvent la principale source de tension avec les récalcitrants. Y avait-il urgence à légiférer sur cette question au milieu d'une session extraordinaire particulièrement chargée ? Je vous en laisserai juges, mes chers collègues. Amenée à se prononcer sur ce texte, notre commission a pris le parti d'adopter une démarche constructive, visant à en améliorer les dispositions au nom de l'intérêt général. La proposition de loi clarifie en effet le cadre législatif de l'interdiction du téléphone portable : à l'autorisation de principe dans l'établissement assortie d'une interdiction absolue dans la classe, l'article 1 substitue une interdiction de principe dans l'établissement, le conseil d'école ou d'établissement pouvant définir des exceptions à cette règle, y compris en classe. J'insiste sur la nécessité, à mes yeux, de renvoyer au conseil d'école ou au conseil d'administration la définition des lieux et des circonstances dans lesquels il peut être dérogé au principe d'interdiction.

Notre commission a considéré que, en clarifiant ainsi le cadre législatif, la proposition de loi donnait une plus grande sécurité aux chefs d'établissement et aux enseignants et permettait d'envoyer un signal fort aux élèves et à leurs parents. J'espère qu'elle participera de la prise de conscience de la nécessité de construire un rapport équilibré aux écrans, en particulier pour les enfants. Les apports de la commission de la culture obéissent à trois principes : cohérence, confiance et simplification. Cohérence, tout d'abord : le champ de la proposition de loi est étendu aux lycées, qui ne sont évidemment pas épargnés pas les difficultés liées à l'utilisation du téléphone portable. Compte tenu de la différence d'âge et de situation, nous avons fait le choix d'un régime, distinct de celui applicable dans le primaire et les collèges. Il s'agit d'une « autorisation d'interdire » donnée au conseil d'administration, ce qui est, vous en conviendrez, particulièrement à propos cinquante ans après mai 68. après mai 68. Confiance envers les chefs d'établissement et les enseignants, ensuite : il s'agit de laisser les établissements libres de fixer les règles les plus appropriées à leur situation particulière, sans les enserrer dans une réglementation bavarde et inutilement précise. C'est en particulier le cas s'agissant de la confiscation des appareils : le texte adopté par l'Assemblée nationale entrait sur ce point dans un luxe de détails inutile et nuisible. Notre commission a entièrement réécrit ces dispositions pour n'en conserver que le principe, renvoyant ses modalités d'application aux établissements, qui sauront adapter leur règlement intérieur en fonction de leur situation. Simplification, enfin : nous supprimons les dispositions non normatives ou ne relevant pas du domaine de la loi, ainsi que les précisions inutiles. Cette proposition de loi somme toute modeste ne doit pas nous exonérer d'un débat plus global sur la place du numérique dans l'éducation et sur l'éducation au numérique, dont la présidente de notre commission, Catherine Morin-Desailly, a rappelé l'urgence dans son récent rapport d'information. Dans son ouvrage, Marcel Gauchet observait qu'« il est impossible à l'école, au risque de se détruire, d'être complètement en phase avec le contemporain. Sa fonction de tradition lui impose d'être toujours en décalage avec les mutations sociales et techniques, ainsi d'ailleurs qu'avec l'événement [ ...]. L'institution scolaire est dans une autre temporalité, faite de rapport au passé, d'anticipation raisonnée du futur, et de lenteur dans l'acquisition des savoirs. Puisse ce texte contribuer à ce que l'école demeure fidèle à sa vocation : qu'elle soit un lieu de concentration, de sociabilité et d'apaisement, où les élèves de notre pays sont mis dans les meilleures conditions pour apprendre et s'élever.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les sénateurs socialistes ont déposé une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, car ils estiment qu'il n'y a pas lieu de légiférer sur ce sujet. N'imaginez pas que le dépôt de cette motion traduise de notre part un excès d'angélisme

Il apparaît néanmoins que ni le législateur ni les responsables des établissements scolaires n'ont attendu cette proposition de loi pour se saisir de la question et pour la régler, généralement de façon simple et efficace. Le code de l'éducation, dans son actuel article L. 511-5, dispose que, « dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite ». Ainsi, toute personne, au fait ou non du droit, constatera-t-elle aisément que le législateur a déjà réglé la question de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire hors lycées, encadrant la réglementation et laissant aux établissements et à leurs conseils d'administration la marge d'autonomie légale pour en régler les détails leur règlement intérieur. Il s'agit d'une solution pragmatique et équilibrée. Quiconque a déjà participé à la vie d'un établissement scolaire, notamment en siégeant dans un conseil d'administration ou dans une commission permanente préparant ces conseils, a eu à se prononcer, à l'occasion de la modification, généralement annuelle, du règlement intérieur, sur la limitation de l'usage des téléphones portables s'appliquant aux élèves au sein de l'établissement concerné. Dans le règlement intérieur des établissements d'enseignement secondaire, on trouve toujours plusieurs lignes prévoyant les lieux et moments auxquels s'applique l'interdiction d'usage de ces appareils et les sanctions dont est passible tout contrevenant.

deuxième exemple d'un règlement intérieur s'applique, cette fois, uniquement dans un collège. Dans la partie « Vivre ensemble », au chapitre consacré aux objets personnels, on lit : « L'utilisation d'un téléphone et de tout type d'appareil audio-vidéo est interdite au sein des bâtiments et durant tous les enseignements les téléphones sont éteints dans les bâtiments. En cas d'utilisation d'un de ces appareils, celui-ci sera retiré à l'élève et sera remis à son responsable légal. » Je précise que, dans ce deuxième cas, le règlement intérieur date de 2013. Deux ans auparavant, en 2011, dans ce même collège, le règlement intérieur portait seulement Le matériel non nécessaire aux études est déconseillé (téléphone portable, lecteur de musique, appareil photographique, etc.) et son utilisation interdite. Je crois avoir apporté la preuve que les établissements savent parfaitement s'organiser et, surtout, qu'ils ont modifié leur règlement intérieur en fonction de l'évolution de l'accès aux technologies et des pratiques des élèves.

et l'introduction de l'article L. 511-5 du code de l'éducation, les chefs d'établissement ont pris conscience des dangers liés à l'usage des téléphones. Ils ont fait voter des mesures de réglementation, voire d'interdiction, de leur usage, dans le cadre des débats qui se déroulent au sein des conseils d'administration et des commissions permanentes, et auxquels participent des représentants de toutes les composantes de la communauté éducative. Je crois donc vous avoir démontré qu'un texte visant à interdire l'utilisation des téléphones au sein des écoles et des collèges et, sur l'initiative de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, à renvoyer aux règlements intérieurs des lycées le soin d'en interdire éventuellement l'usage, ne sert à rien, sinon à entamer l'autonomie des établissements voulue par les lois de décentralisation, ainsi que le pouvoir délibératif des organes internes des établissements et l'autorité des chefs d'établissement.

Loin de simplifier la tâche des établissements, ce nouveau dispositif inverse la logique qui prévalait pour fonder les interdictions et va complexifier la mise en place de règles claires l'utilisation du téléphone ne sera plus interdite où et quand le règlement le prévoira mais sera, au contraire, permise où et quand le règlement le prévoira. Il est toujours beaucoup plus compliqué de prévoir des exceptions que d'établir une interdiction claire ! Je suis d'autant plus étonnée par cette proposition de loi que, à ma connaissance- j'ai entendu nombre de représentants des membres de la communauté éducative -, ni le syndicat majoritaire des personnels de direction ni les représentants des parents d'élèves n'étaient demandeurs d'une telle modification législative ... Seule l'extension aux lycées de l'actuel dispositif de l'article L. 511-5 du code de l'éducation,

On demande une fois de plus au Parlement de servir de caution à la communication du Gouvernement et à sa majorité ! Le message transmis est incomplet, et donc malhonnête. Je m'étonne également de la démagogie dont a fait preuve la majorité de l'Assemblée nationale. Sans doute conscients que le dispositif de la proposition de loi était fort contestable, les députés ont souhaité compléter le texte par plusieurs articles additionnels pour- prétendument -renforcer l'éducation à l'utilisation d'internet et des outils numériques. Néanmoins, l'un des articles du code de l'éducation que les députés se proposaient de compléter au travers de l'article 2 était de portée bien trop générale pour qu'il y soit fait mention de l'éducation à « l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne ». Sur proposition de notre rapporteur, il a fort heureusement été supprimé en commission. Les deux autres articles ajoutés ne bouleversent en rien l'arsenal déjà prévu par le code de l'éducation pour sensibiliser les élèves et les étudiants aux dangers de l'internet.

d'une utilisation « responsable » de ces outils ou substituer à la « sensibilisation » une « éducation » aux droits et devoirs liés à l'usage d'internet et des réseaux ne révolutionnera en rien l'éducation à l'utilisation des outils d'internet et aux droits et devoirs de l'internaute. De telles modifications prêteraient presque à sourire si elles ne figuraient pas dans le texte On ne pourra également que s'étonner de la précision figurant à l'article 4, selon laquelle les projets d'école et d'établissement pourront prévoir des expérimentations sur « l'utilisation des outils et ressources numériques la nature législative d'une telle disposition n'est pas avérée et, dans la pratique, les projets d'école et d'établissement sont déjà très souvent axés autour de cette utilisation. Ces articles introduits par l'Assemblée nationale, de portée normative extrêmement limitée, permettront vraisemblablement au législateur de se donner bonne conscience

Rien ne justifiait de demander au Parlement de travailler sur un problème certes très important, mais dont les solutions résident non pas dans la mise en oeuvre d'une nouvelle loi, mais dans une application plus stricte de la loi actuelle et dans un renforcement de l'éducation parentale et de la pédagogie scolaire. Toutes ces raisons nous conduisent à considérer qu'il n'y a pas lieu de débattre sur la proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, et à demander au Sénat de bien vouloir adopter notre motion tendant à opposer la question préalable.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a maintenant plus d'un demi-siècle, les récepteurs de télévision entraient progressivement dans les foyers français. Ils allaient bien souvent y bouleverser les habitudes. Ces profonds changements semblent aujourd'hui pourtant bien modestes à côté de celui que représente, depuis plus d'une décennie, l'omniprésence, tant au sein du foyer qu'en dehors, d'internet et des supports d'utilisation mobiles qui l'accompagnent.

Au-delà de son aspect utile et ludique, cette pratique est clairement addictive et, comme pour toute pratique addictive, nous avons un devoir de vigilance tout particulier à l'égard de nos enfants.

ces appareils est source de repli sur soi à un âge où nos adolescents ont déjà une tendance à l'isolement. Certains jeunes s'enferment de fait dans un espace où la parole des adultes, habituellement source de modération, est exclue et où seule la parole adolescente a droit de cité. Par le biais des réseaux sociaux, ils se trouvent ainsi exposés à des formes de harcèlement particulièrement dévastatrices. Alors que le temps scolaire devrait justement permettre de rompre cet isolement et de porter le plus efficacement possible la parole des adultes, l'usage du smartphone vient contrarier ce nécessaire dialogue intergénérationnel.

à dégrader la qualité du climat scolaire, la présence du téléphone portable dans nos écoles, collèges et lycées soulève aussi un enjeu pédagogique. Incontestable facteur de dispersion, leur utilisation récurrente en classe conduit les enseignants à consacrer à la discipline un temps qui ne profite pas à l'instruction. profite pas à l'instruction. On constate aisément que l'interdiction des téléphones portables au sein des enceintes scolaires s'accompagne généralement d'un regain de concentration et d'une amélioration des résultats, notamment chez les élèves les plus en difficulté. Cette nécessité d'agir, la communauté éducative en a pris conscience depuis longtemps. Un grand nombre de collèges interdisent déjà leur règlement intérieur l'usage d'un téléphone mobile en classe.

En effet, en dehors de la classe, la libre utilisation demeure la règle, et les interdictions étendues à l'ensemble des enceintes scolaires présentent une fragilité juridique. En outre, la confiscation fait également aujourd'hui l'objet d'interprétations diverses. diverses. Les circulaires ministérielles n'en font mention que dans le cas d'objets toxiques ou dangereux. Enfin, les dispositions actuelles ne permettent pas l'utilisation des téléphones portables multifonctions dans un cadre pédagogique en classe. après avoir procédé à l'équipement des élèves en outils numériques, avec des résultats mitigés, nos collectivités territoriales privilégient aujourd'hui l'utilisation d'un matériel appartenant déjà aux élèves.

Si nous partageons également la volonté de nos collègues de préserver l'autonomie de la communauté éducative, qui demeure la mieux à même d'évaluer et de faire évoluer ses règles de fonctionnement, nous sommes convaincus que celle-ci est aujourd'hui dans l'attente d'un cadre plus sécurisant. Sur la forme, comme beaucoup de nos collègues, nous nous montrerons beaucoup plus réservés. Le Gouvernement et sa majorité ont choisi la voie législative pour mener à bien cette réforme. D'autres démarches auraient sans doute pu permettre de parvenir à un résultat identique, même s'il faut bien reconnaître les lacunes de l'article L. 511-5 du code de l'éducation. Le calendrier retenu pour l'examen de la présente proposition de loi prête aussi à interrogations, alors que les textes d'envergure se succèdent. Nous sommes nombreux à penser que le temps parlementaire pourrait être mieux utilisé.

En dépit de ces réserves sur la forme, nous adhérons aux propositions qui nous sont faites par la commission de la culture du Sénat. L'éducation dans le cadre scolaire suppose aussi d'apprendre à nos enfants à vivre sans écran. L'univers numérique évoluant vite, il est fort probable que de nouvelles adaptations seront prochainement à envisager, sans que celles-ci aient d'ailleurs nécessairement à faire de nouveau l'objet d'une loi.

Cette réflexion, le Sénat s'emploie déjà à la mener à travers les travaux de Mme la présidente de la commission de la culture, qui a récemment produit un rapport rappelant l'impérieuse nécessité de la formation pour prendre en main notre destin numérique.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à encadrer l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires. sein de notre commission de la culture, le changement de paradigme proposé par les auteurs de ce texte, substituant au régime actuel d'autorisation un régime d'interdiction assorti d'exceptions, a suscité un certain scepticisme quant à l'utilité de légiférer. Nous devons pourtant bien admettre deux réalités. La première, c'est que nous sommes tous d'accord ici sur le fond, à savoir le bien-fondé de l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable par les élèves dans les établissements scolaires. Je crois même que certaines divergences proviennent d'une vive inquiétude unanimement partagée, mais exprimée de manière différente. En effet, au-delà du cas de nos enfants, ce texte pousse chacun d'entre nous à s'interroger sur l'usage des téléphones portables dans notre vie quotidienne, sur leur omniprésence dans nos sphères professionnelle, personnelle

voire inquiétante, surtout lorsque nous voyons nos enfants et nos petits-enfants s'emparer de cette technologie avec une aisance déconcertante, parfois abusivement, souvent sans précautions. Dans ces conditions, lorsqu'il est question d'encadrer l'utilisation des téléphones portables dans l'enceinte de l'école, pilier sacré de notre pacte républicain, le sujet devient encore plus sensible, tant nous savons qu'il est de notre responsabilité d'apprendre à nos enfants à maîtriser l'usage de cet outil exceptionnel. La seconde réalité, c'est que le cadre juridique actuel est défaillant. S'il a permis la mise en place de bonnes pratiques dans certains établissements, nous ne pouvons pas nier qu'il en existe aussi de très mauvaises. Très concrètement, la loi ne permet pas aujourd'hui d'interdire le téléphone portable dans l'ensemble de l'enceinte de l'établissement, le principe de liberté d'utilisation en dehors de la classe demeurant la règle. Or nous savons que le téléphone induit des risques qui vont bien au-delà de la triche ou du déficit de concentration en classe, depuis les vols ou le racket jusqu'au cyberharcèlement et au visionnage de contenus violents ou inadaptés : autant de risques dont l'école doit protéger nos enfants lorsqu'ils sont dans ses murs. Je ne m'étendrai pas sur les effets bénéfiques d'un meilleur encadrement. Le premier enjeu est évidemment celui de l'assiduité des élèves et son corollaire, le climat scolaire. Le second enjeu est de santé publique, tant on sait qu'un usage intensif des téléphones portables, et plus largement des écrans, peut engendrer des problèmes relationnels et émotionnels, des troubles du sommeil ou encore des phénomènes de dépendance et d'addiction. Cela étant dit, j'entends naturellement, sans vraiment les comprendre, les voix qui s'élèvent pour dénoncer une mesure de communication, inutile pour certains, inopérante pour d'autres. Nous savons bien que ce texte ne répondra pas à la grande complexité d'un tel sujet de société, mais devons-nous, pour autant, le balayer d'un revers de main Pourquoi ne pas y voir au contraire une occasion d'apporter une pierre supplémentaire, aussi modeste soit-elle, à l'édifice de notre école républicaine, de manière à la rendre plus forte, plus protectrice ? la situation de défaillance que j'ai décrite impose non seulement de faire évoluer les dispositions actuelles, mais de le faire par la loi, avec ses vertus tant juridiques que symboliques. En encadrant l'usage du portable dans les écoles et les établissements, c'est aussi un signal que nous enverrons : cela montrera que nous légiférons dans le concret pour mieux sensibiliser les élèves et les familles aux usages raisonnés des écrans.

Je partage également son attachement aux dispositions prévoyant la formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques et le développement de l'esprit critique, ainsi qu'une véritable éducation aux droits et devoirs liés à l'usage d'internet. Dans cet esprit, je proposerai de rétablir, à l'article 1, la précision selon laquelle l'interdiction ne s'applique pas aux usages pédagogiques. S'il est sous-entendu que chaque établissement prendra en compte cet aspect dans son règlement intérieur, je considère qu'il est important que la loi l'assume explicitement. enseigné pendant de très longues années, j'ai souvent entendu le refrain selon lequel les livres, le papier resteraient de meilleurs supports d'enseignement que les nouvelles technologies.

jeunes à utiliser ces outils avec discernement, c'est-à-dire encourager les bons usages et empêcher les mauvais, c'est bien la manière la plus volontariste, pour l'école, de relever les défis de la révolution numérique en cours. Fort de ces réflexions et bien conscient que ces dispositions ne prendront leur pleine mesure qu'à l'épreuve du terrain, notre groupe votera en faveur de l'adoption de cette proposition de loi

pour les institutions de l'Ancien Régime, une procédure par laquelle le souverain pouvait imposer sa décision au Parlement. Celui-ci perdait alors son pouvoir discrétionnaire pour ne plus être qu'une chambre d'enregistrement, selon l'adage- quand le Prince vient, le magistrat quand le Prince vient, le magistrat s'interrompt. À lire le texte de la rapporteur de l'Assemblée nationale sur cette proposition de loi, celui de son collègue président de la commission de la culture et des députés de leur majorité, on peut se demander si sa première et seule légitimation ne réside pas dans l'obligation acceptée de satisfaire, selon la même sentence, un engagement pris par le Président de la République à l'occasion de sa campagne.

l'objectif est que cette réforme s'applique à partir de la rentrée scolaire de 2018 sous réserve, bien évidemment, du déroulement de nos débats à l'Assemblée, puis au Sénat.

Nous comprenons bien ici que cette forme de servitude volontaire exprime l'inclinaison vers laquelle est entraînée la réforme constitutionnelle en cours. La proposition de loi est l'instrument de l'initiative parlementaire en matière législative. En l'occurrence, l'Assemblée nationale l'a mise à disposition de l'expression de la volonté présidentielle. Nous savons gré à notre collègue députée de nous laisser encore la liberté de maîtriser le déroulement de nos débats. En revanche, je m'associe aux remerciements adressés à notre collègue Stéphane Piednoir, qui a tenté de faire la part des choses et de donner un peu de substance juridique à un texte qui en était singulièrement dépourvu. Qu'on en juge ! L'article L. 511-5 du code de l'éducation dispose que « dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite ». Cette rédaction sans ambiguïté marque une interdiction générale de l'utilisation du téléphone dans les établissements cités, tout en laissant la possibilité aux équipes pédagogiques de définir, par le biais du règlement intérieur, les lieux où elle ne s'exercerait pas. La nouvelle rédaction proposée pour cet article n'apporte aucune extension ou confortation juridique majeure au dispositif actuel. Ses seules plus-values sont l'ajout de la notion d'« équipement terminal de communications électroniques » à celle de « téléphone mobile », la mention explicite dans la loi de la possibilité d'interdire ces équipements dans les lycées par le biais des règlements intérieurs et de pouvoir en autoriser la confiscation de la même façon.

Dans la pratique, aucun exemple ne nous est rapporté de situations dans lesquelles l'actuel dispositif de l'article L. 511-5 du code de l'éducation se serait révélé inapproprié ou aurait placé les équipes pédagogiques dans des situations de fragilité juridique. Bien au contraire, il aurait été précieux de dresser un bilan des expériences nombreuses ayant permis aux enseignants, dans nombre d'établissements, de mettre à profit la discussion collective sur le règlement intérieur pour engager un débat très utile, avec les élèves et leurs parents, sur les conditions d'utilisation des Pourquoi faudrait-il absolument valider par la loi les bonnes pratiques locales, alors qu'il suffirait de leur donner la publicité qu'elles méritent pour en favoriser la diffusion ? La vérité ne procéderait-elle que du haut vers le bas ? Effaré par la minceur du sujet de cette proposition de loi, je me suis finalement demandé, comme notre collègue Antoine Karam, si son objet inconscient n'était pas de soigner un mal-être général et d'exiger de l'enfant

car il ne faudrait pas que ces ratiocinations nous le fassent oublier, il est urgent d'ouvrir un vaste chantier de recensement, d'évaluation et de confrontation des expériences foisonnantes réalisées dans l'utilisation du numérique pour l'enseignement. Forte de son indépendance, de ses compétences reconnues dans ce domaine et de son esprit constructif, la Haute Assemblée est à votre disposition, monsieur le ministre, pour engager avec tous les acteurs la réflexion générale sur ces sujets ; c'est peut-être

À l'heure où se prépare l'évolution de notre Constitution, se pose une fois de plus la question de l'articulation entre la loi et le règlement. Pour appuyer le paradoxe de la situation, rappelons que la réforme du baccalauréat est, elle, d'ordre réglementaire. Nous n'aurons donc pas- hélas ! -l'occasion d'en débattre dans cette enceinte. Pourtant, quel sujet majeur ! majeur ! Le texte que nous discutons n'en a pas moins une valeur symbolique importante, puisqu'il rappelle qu'il y a des règles à l'école. Exactement ! Au travers de cette question de l'usage du téléphone portable, il s'agit bien ici de remettre en évidence la nécessaire organisation de l'autorité à l'école et le rôle tenu par l'éducation nationale et ses représentants,

peut accentuer l'incapacité de certains élèves à se concentrer et à se structurer. Mais on sait aussi que de plus en plus d'établissements et d'enseignants ont pris possession de l'outil numérique dans le cadre des cours. Il faut donc encadrer, mais avec discernement.

Pour aller plus au fond du texte, on sait que le cadre législatif actuel est incertain et inadapté. Si un nombre élevé d'établissements scolaires pratiquent une interdiction totale du téléphone portable, c'est en l'absence de cadre juridique adapté. adapté. Le code de l'éducation dispose actuellement que « dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite La modification législative qu'il nous est proposé d'adopter s'inscrirait dans un projet éducatif précis et encadré par le personnel éducatif. La voie législative est, d'ailleurs, l'option juridique la plus sûre pour garantir l'effectivité de l'interdiction des téléphones portables.

Ce n'est pas notre présidente de la commission de la culture, Mme Catherine Morin-Desailly, qui a de nombreux éclairages à nous fournir sur le sujet, qui dira le contraire ! L'école du XXI siècle doit former au numérique, en le prenant comme outil d'apprentissage et instrument de vie, qu'il faut savoir manier avec discernement.

Nous pouvons nous féliciter que le rapporteur, Stéphane Piednoir, ait retiré du texte des précisions qui transformaient véritablement le code de l'éducation en règlement intérieur d'établissement. Dans un souci de cohérence et d'exhaustivité, les membres de la commission de la culture ont donc étendu le champ de la proposition de loi aux lycées, en prévoyant un régime d'encadrement spécifique, distinct du régime défini pour les écoles et les collèges. Afin de sécuriser la pratique de la confiscation et dans le respect de l'autonomie des établissements, ils ont par ailleurs récrit les dispositions relatives à la confiscation, notamment en étendant la faculté d'y procéder aux personnels d'éducation et de surveillance. Privilégiant l'autonomie des établissements et l'appropriation de la règle par l'ensemble de la communauté éducative, ils ont supprimé les précisions inutiles qui affaiblissaient le rôle du règlement intérieur. Enfin, fidèle aux orientations du Sénat en matière de qualité de la loi, la commission de la culture a supprimé plusieurs dispositions inutiles ou superfétatoires, dont celles

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous avons à examiner aujourd'hui a été accueillie par nombre d'entre nous avec une certaine circonspection. Il s'agit, certes, d'une promesse de campagne du Président de la République et il n'est jamais de bon ton de critiquer la volonté de respecter ses engagements, de mettre en accord ses discours et ses actes.

L'article L. 511-5 du code de l'éducation dispose ainsi que, « dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite ». S'agit-il d'élargir la notion de téléphone mobile pour inclure les appareils électroniques qui n'existaient pas à l'époque élément oublié dans la rédaction initiale. S'agit-il de revenir sur la souplesse qu'offre le cadre des règlements intérieurs des établissements scolaires ? Le Gouvernement ne fait malheureusement pas la démonstration de l'irrépressible nécessité de rogner ainsi l'autonomie des établissements scolaires, jetant une pierre supplémentaire dans le jardin de la décentralisation,

Peut-être s'agit-il, plus prosaïquement, de la simple volonté d'effectuer une opération de communication politique, au risque d'engendrer une charge administrative supplémentaire ?

risque de provoquer une inflation des règlements intérieurs, sans parler de la nécessité de prendre en compte l'ensemble des situations susceptibles de permettre un usage encadré de ces dispositifs électroniques. Je suis bien plus enclin à accorder ma confiance à la capacité d'initiative des communautés éducatives des établissements, permettant une mise en oeuvre contextualisée de l'encadrement de l'usage des dispositifs de communication électronique. Par exemple, concernant les règles de saisie des appareils, chaque établissement peut actuellement définir sa politique au regard des considérations locales. Pourquoi priver les acteurs de terrain de leur capacité d'adaptation ?

Le Gouvernement serait-il dans l'obligation de se prévaloir de l'instauration de nouvelles dispositions à chaque rentrée scolaire ? Cette proposition de loi, au mieux, n'ajoute rien à l'existant ; au pire, elle risque de complexifier les tâches de régulation au sein des établissements.

Je ne peux que saluer la suppression, sur l'initiative du rapporteur, de l'article 2, dont le mérite principal était de creuser encore un peu plus le sillon, décidément fertile, des déclarations de principe sans portée normative, alimentant avec allégresse l'inflation législative. De même, la suppression, à l'article 3, de l'expression « citoyenneté numérique » est une bonne chose, le concept semblant pour le moins évasif, voire problématique. L'apprentissage de la citoyenneté apparaît en effet comme un ensemble cohérent, auquel il ne semble pas nécessaire d'adjoindre des qualificatifs, sauf à estimer que l'on pourrait encourager l'apprentissage des comportements citoyens dans certaines circonstances ou dans certains espaces, et pas dans d'autres. Nous sommes tous conscients des enjeux inhérents à la diffusion massive des téléphones « intelligents » et des dérives qu'une pratique irraisonnée peut engendrer

C'est une situation sans précédent, dont les effets débordent très largement le cadre strictement scolaire et interrogent l'évolution de notre société. Les dérives dans l'usage de ces appareils technologiques ne doivent pas atteindre l'enceinte éducative. C'est néanmoins parfois le cas, et la modification législative aujourd'hui soumise à notre examen semble s'égarer dans une forme de discours performatif. Mais, en l'occurrence, dire n'est pas faire pas faire ! On ne voit pas en quoi ce texte et les changements qu'il tend à opérer sont de nature à faciliter la mise en oeuvre de la régulation de l'usage de ces appareils électroniques. Le renversement de la logique vers une interdiction générale assortie d'exceptions ne remédiera pas, comme par enchantement, à l'existence de situations potentiellement conflictuelles. Les difficultés d'application des règles, rencontrées avec certains élèves, voire parents d'élèves, récalcitrants, militent très nettement pour le maintien d'une gestion décentralisée de ces situations. Cela manifesterait, en outre, la confiance placée dans les équipes de chaque établissement au regard de leur capacité à faire vivre et à appliquer concrètement ces principes. L'absence de réflexion en amont sur le sujet plus vaste de l'éducation au numérique et de l'usage responsable des nouvelles technologies est regrettable, d'autant que Mme la présidente de la commission sénatoriale de la culture, de l'éducation et de la communication vient de présenter un excellent rapport sur cette question. L'Assemblée nationale elle-même travaille sur le thème de l'école dans la société du numérique. Les dispositions de cette proposition de loi auraient certainement été bien plus utilement discutées et travaillées dans le cadre d'une initiative législative plus large, permettant d'appréhender toutes les dimensions de la question.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au travers de l'examen de cette proposition de loi, nous sommes invités à nous prononcer sur notre vision de l'éducation à l'ère du numérique.

dans les établissements scolaires, tout en ouvrant la voie à des autorisations possibles, il offre une clarification juridique salutaire et pose, pour reprendre les propos de Mounir Mahjoubi, des « règles pour éviter le pire ». Les deux plus grandes figures du numérique, Bill Gates et Steve Jobs, avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. En 2007, l'ancien PDG de Microsoft avait lui-même instauré une durée limitée d'exposition aux écrans pour ses enfants et leur interdisait l'usage d'un téléphone portable avant l'âge de quatorze ans. Pour le reste de la société, l'âge moyen de possession d'un premier téléphone est de dix ans. Tous les enfants ne sont pas égaux face aux risques que représente l'usage incontrôlé des nouvelles technologies ... « J'échangerai toute ma technologie pour un après-midi avec Socrate », disait pour sa part Steve Jobs. Nous connaissons déjà les risques, pour les enfants, d'une exposition excessive aux écrans troubles de l'attention et du comportement, myopie, troubles de l'apprentissage, risques d'exposition aux contenus violents ou pornographiques, cyberharcèlement La liste est longue, et les jeunes victimes de harcèlement les réseaux sociaux sont nombreuses. L'école doit rester un sanctuaire ! Nous savons également que les risques de dépression augmentent pour un adolescent avec la fréquentation des réseaux sociaux. Le recul de l'exercice physique et la diminution du temps de lecture sont aussi des effets collatéraux de la dépendance des enfants aux écrans. la London School of Economics a démontré que les résultats scolaires progressaient après l'application d'une interdiction des téléphones portables dans les écoles. Aussi cette proposition de loi nous apparaît-elle à tout point de vue bénéfique pour préserver l'équilibre des élèves et la qualité de l'apprentissage. Je me félicite de l'adoption Je me félicite de l'adoption en commission d'un amendement visant à laisser à l'établissement la liberté de définir le mode de restitution de l'objet confisqué. J'avais moi-même déposé un amendement allant dans ce sens. Pour autant, l'utilisation des téléphones et des tablettes à des fins pédagogiques reste possible. Je pense, d'ailleurs, que le numérique est la voie de prédilection vers l'auto-apprentissage et offre des possibilités d'enseignement illimitées Ainsi, aux États-Unis, la plateforme dématérialisée HarvardX met à disposition du monde entier des cours de très haut niveau. Les possibilités de partenariats internationaux, d'échanges de pratiques et de savoirs sont démultipliées avec le numérique. À ce titre, le rapport intitulé « Vers une société apprenante », remis par François Taddei en avril dernier, préconise la mise en place d'un campus national numérique pour fédérer les apports de chaque établissement d'enseignement. Pour limiter les effets néfastes sur les enfants de l'exposition aux écrans dans le cadre des activités pédagogiques, je défendrai un amendement visant à équiper les écrans utilisés par les élèves de filtres à lumière bleue.

L'adoption de cette proposition de loi sera une première étape vers un équilibre qu'il reste à trouver entre développement technologique et capacité de la société à en faire bon usage. Aussi, au-delà du texte en lui-même, il s'agira de veiller à sensibiliser l'ensemble de la société à une utilisation maîtrisée des outils numériques,

Le téléphone portable ne sert plus uniquement à téléphoner. Une multitude d'usages se sont développés : navigation sur internet, prise de photos, réalisation de films, visionnage de vidéos, jeux et, bien sûr, échange de messages. Ces smartphones soulèvent donc des enjeux pédagogiques et disciplinaires, tout particulièrement au collège, mais pas la possession de ces outils de communication est de plus en plus fréquente dès l'école élémentaire, ce qui me semble particulièrement inquiétant. Le climat scolaire s'en trouve trop souvent altéré. Plusieurs raisons m'amènent à me prononcer en faveur de l'interdiction des téléphones dans les écoles et collèges. Les téléphones portables, tout comme les vêtements, peuvent affirmer des disparités sociales entre enfants. À l'instar de l'initiative prise par certains établissements d'instaurer des tenues obligatoires afin de gommer ces différences, je suis favorable à l'interdiction de ces appareils, pouvant être perçus comme des signes extérieurs de richesse, susceptibles de créer un climat de comparaison malsain et frustrant entre camarades.

en détient un. Racket et responsabilité en cas de détérioration risquent de causer des problèmes dont la communauté éducative, les enfants et les parents d'élèves se passeraient bien volontiers. ailleurs, l'utilisation du portable pendant les cours porte atteinte à la capacité d'attention et de concentration des élèves. Elle conduit à une dispersion peu propice à la réflexion, à la compréhension et à la mémorisation des enseignements. outre, elle peut favoriser la paresse- les élèves ne cherchant plus les réponses dans leurs connaissances personnelles -, le plagiat et, bien sûr, la « triche » lors des contrôles. La nouvelle génération dispose d'un accès facilité aux réseaux sociaux sans avoir forcément une maîtrise intelligente de ces nouvelles technologies.

chez les élèves en grande difficulté. Ses auteurs ont conclu que la limitation de l'usage du téléphone portable à l'école pouvait constituer un moyen de réduire les inégalités dans l'éducation.

Les effets des radiofréquences sur la santé des enfants restent mal connus, mais, dans un rapport de 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a déjà souligné que les enfants pouvaient être plus exposés à ces radiofréquences que les adultes, en raison de leurs spécificités morphologiques, anatomiques et physiologiques.

visionnage d'un contenu inadapté à un public jeune auquel les enfants pourraient avoir accès en naviguant sur internet hors du contrôle d'un adulte. Il me semble donc judicieux que l'institution scolaire se fasse un devoir de contrôler l'usage du téléphone lorsque les enfants se trouvent sous sa responsabilité.

L'école est là pour donner l'exemple aux enfants, mais aussi aux parents. Bien souvent, la prévention assurée dans le cadre scolaire produit ses effets au-delà de l'école et s'étend au cercle familial par la voix de l'enfant.

Ces précisions étaient, de mon point de vue, nécessaires, car, monsieur le ministre, ce n'est pas à un juriste comme vous qu'il faut rappeler l'adage romain :. Quand les lois sont trop nombreuses, elles perdent en qualité. Fallait-il avoir recours à un tel arsenal législatif quand une circulaire aurait pu suffire ? Les sanctions en cas d'infraction à la loi ne créeront-elles pas des lourdeurs nouvelles et des contentieux inutiles dans ce qui touche à l'éducatif, au pédagogique, à la vie scolaire ? Je ne vous cache pas que je m'interroge Je sais toutefois que notre droit positif prévoit déjà, depuis la loi de 2010 portant engagement national pour l'environnement, une telle interdiction pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que pour les collégiens. Je ne souhaite pas polémiquer sur la portée concrète de cette interdiction ni entrer dans une opposition stérile. Espérons que cette discussion parlementaire servira à sensibiliser les familles sur les conséquences d'un usage excessif ou inapproprié du téléphone portable par les enfants et les adolescents.

Nos jeunes sont donc de plus en plus exposés aux écrans. Cette situation n'est pas sans conséquence. De nombreuses études l'ont montré, qu'elles émanent de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l'Académie des sciences ou de professionnels de santé reconnus. Toutes pointent les effets désastreux de la surexposition aux écrans : troubles du sommeil, de l'attention, voire difficultés cognitives ou état dépressif. Nous sommes ici pour nous interroger sur les risques liés à une exposition à des contenus inappropriés dans l'enceinte des établissements scolaires, notamment à l'heure de la récréation et lors de la pause méridienne. En effet, il est à craindre que ces temps partagés puissent être l'occasion d'émulations malsaines liées à des phénomènes de groupe. de vidéos pornographiques librement accessibles sur les plateformes de téléchargement et de, de sites véhiculant des thèses complotistes, de blogs communautaristes incitant à la violence religieuse et propageant la haine antisémite la plus virulente, ou encore au cyberharcèlement, qui, bien souvent, se prolonge au domicile, ne laissant aucun Dans son récent rapport d'information consacré à la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, notre collègue Marie Mercier relève que, dans un contexte d'hypersexualisation les smartphones, on constate de plus en plus « « le développement de comportements sexuels de la part de jeunes enfants, parfois de très jeunes enfants, qui tentent de reproduire entre mineurs des scènes pornographiques, de plus en plus " extrêmes " ». Oui, mes chers collègues, il est nécessaire de réfléchir à l'usage des terminaux connectés, aux contenus accessibles et aux effets d'une surexposition aux écrans pour les plus jeunes, que ce soit pendant le temps scolaire ou en dehors. Je soutiendrai donc toute initiative qui contribuera à protéger nos élèves. Même si la loi ne me paraît pas être le véhicule le plus souple, l'intention des auteurs

des tyrannies de l'instant. En effet, si l'école est un lieu de transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, elle est aussi un lieu de prise de distance par rapport au quotidien, au bruit de la rue, une sorte de sanctuaire laïque et républicain.

Pourtant, il a semblé à nos collègues députés que les seuls règlements intérieurs des établissements n'avaient pas une portée suffisante et qu'il était nécessaire de s'appuyer sur un cadre plus sécurisé. Pour autant, mes chers collègues, monsieur le ministre, légiférer était-il nécessaire ?

dubitatif quant à l'intérêt d'en passer par la loi. Je m'associe pourtant volontiers à cette démarche, qui envoie un signal d'ordre à une école pouvant apparaître parfois confrontée à une crise d'autorité. Je veux donc saluer les apports de notre collègue Stéphane Piednoir, qui ont permis de renforcer la cohérence de ce texte. Je pense à l'introduction d'un régime particulier pour les lycées ou à la suppression de mesures bavardes, détaillant par exemple les procédures de confiscation. Toutefois, monsieur le ministre, mes plus vives interrogations portent sur l'intérêt de débattre quelques heures sur ce sujet alors que tant de grandes réformes que vous portez, avec un réel succès d'ailleurs, ne donneront pas lieu à une seule heure d'échanges dans cet hémicycle. Je veux parler, notamment, de la réforme du baccalauréat, de ses effets sur la réorganisation des lycées ou de la rénovation de la voie professionnelle.

Il est vrai que la révolution numérique transforme l'accès à la connaissance, interroge comme jamais le métier de professeur, bouscule le rapport maître-élève, oblige à repenser la formation initiale des enseignants et rend nécessaire la relance de la formation continue. C'est de ces sujets, monsieur le ministre, que nous espérons pouvoir un jour débattre, car nous sommes persuadés que vous avez beaucoup de choses à nous dire et un cap à fixer.

Cela a été rappelé, l'usage du téléphone portable en classe est déjà réglementé, au moins durant toute la durée des enseignements, mais tout le monde fait le constat des dégâts qu'il provoque : problèmes relationnels, troubles de la concentration et de la mémorisation, troubles des apprentissages. Tout cela rend la classe et le milieu scolaire invivables. Nous pouvons tous observer le spectacle affligeant de ce que sont devenues les cours de création du fait de l'omniprésence du portable.

l'enseignement. L'école doit être par excellence le lieu de la déconnexion. C'est à l'écart et à l'abri d'internet que peuvent se former les élèves. Ils ont besoin d'être soustraits au monde environnant, à son agitation, à son brouhaha.

a pu avoir un sens, ce n'est plus le cas aujourd'hui, tant les outils numériques font partie du quotidien de chacun. Il est nécessaire de former les jeunes à leur usage et de considérer les plus-values qu'ils apportent Ainsi, autoriser l'usage des appareils électroniques dans un cadre pédagogique permettrait d'inscrire dans la loi le renforcement de l'éducation des jeunes au regard des enjeux numériques, en vue de les responsabiliser et de les former aux nouvelles technologies. Cela a été dit,

portant engagement national pour l'environnement ; prévoir que l'utilisation d'un téléphone portable en méconnaissance des règles fixées à cet article ne peut entraîner sa confiscation que si cette sanction est prévue par le règlement intérieur. Pour justifier le rétablissement de l'article L. 511-5 du code de l'éducation, les auteurs de l'amendement soutiennent que la quasi-intégralité des établissements interdiraient déjà l'utilisation du téléphone portable dans leurs locaux. L'objet de la proposition de loi est justement de sécuriser ces interdictions, dont la légalité pourrait être contestée, dès lors que si le règlement intérieur peut évidemment encadrer l'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte des établissements scolaires, il ne peut pas, en revanche, édicter une interdiction générale et absolue. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite que le principe de l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable s'impose dans toutes les écoles et dans tous les collèges, sans qu'il faille s'en remettre à la volonté de l'autorité chargée d'adopter le règlement intérieur, à savoir le conseil d'école ou le conseil d'administration pour les collèges. Ces derniers pourront néanmoins décider, le cas échéant, des lieux et des circonstances dans lesquels l'utilisation du téléphone portable pourrait éventuellement être autorisée. Les auteurs de l'amendement entendent par ailleurs sécuriser le droit à la confiscation d'un téléphone portable en précisant que cette sanction ne peut intervenir que si elle est prévue par le règlement intérieur. Or l'objet de la proposition de loi n'est pas d'ériger la confiscation du téléphone portable en sanction disciplinaire, au sens de l'article R.511-13 du code de l'éducation. La confiscation représente en l'espèce une simple punition scolaire, constitutive d'une mesure d'ordre intérieur, qui peut être décidée par tout personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance de l'établissement. Dans ces conditions, il semble plus adapté de renvoyer au règlement intérieur le soin de préciser les modalités concrètes de sa mise en oeuvre- durée, information des parents, restitution -, plutôt que de les inscrire dans la loi. La confiscation de l'appareil ne fera par ailleurs pas obstacle, dès lors qu'il s'agit, comme cela a été dit, d'une simple punition, et non d'une sanction disciplinaire, à l'engagement d'une procédure disciplinaire susceptible d'aboutir au prononcé d'une des sanctions prévues à l'article R.511-13 lorsque les circonstances le justifieront, par exemple en cas de récidive ou d'utilisation portant atteinte à l'image et à la dignité d'un élève ou d'un membre de la communauté éducative. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l'amendement n° 4. L'amendement n° 7 a pour objet de rétablir une exception au principe général d'interdiction de l'usage du téléphone portable.

à des fins pédagogiques au regard des évolutions technologiques que connaît la société. Ces usages pédagogiques doivent être encadrés, construits par les enseignants dans le cadre de démarches pédagogiques au service de l'apprentissage des élèves. C'est une des vertus de cette proposition de loi que d'être beaucoup plus explicite sur la question. Il s'agit de faciliter le travail des équipes de direction et des enseignants, en leur donnant un point d'appui législatif, un repère clair et une base juridique solide. Nombre d'écoles et d'établissements d'enseignement scolaire ont mené

Toutefois, il s'agit là de démarches pédagogiques qui doivent être strictement encadrées, et c'est donc uniquement sous l'autorité du professeur que cela peut se concevoir. Enfin, le Gouvernement souhaite non seulement ne pas remettre en cause ces expérimentations, mais aussi les encourager, dès lors dès lors qu'elles permettent d'associer les représentants de la communauté éducative. Pour l'ensemble de ces raisons, je suis favorable à l'amendement n° 7. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

tablettes et ordinateurs utilisés dans le cadre des activités pédagogiques. Les écrans sont devenus la première occupation des enfants et adolescents. Scientifiques et professionnels ont alerté les parents et les pouvoirs publics sur les effets néfastes, pour la santé et le développement de l'enfant, de la surexposition aux écrans retard dans l'acquisition du langage, troubles de l'attention, désorientation du regard, troubles relationnels, troubles du sommeil et myopie. Par ailleurs, une étude PISA datant de 2015 a montré que les enfants utilisant le moins les outils numériques dans le cadre scolaire en font meilleur usage, car ils ont pu développer au préalable des capacités de synthèse et de hiérarchisation de l'information. Quel est l'avis de la commission ? Madame Mélot,

Il ne paraît pas utile de graver dans la loi de telles dispositions, à plus forte raison lorsqu'il est fait référence à des notions scientifiques, qui, par nature, peuvent évoluer dans le temps.

: La parole est à Mme Colette Mélot. Cet amendement vise à protéger les enfants de l'exposition à la lumière bleue des écrans utilisés à des fins pédagogiques ou pour des raisons de santé ou de handicap, pendant le temps scolaire. de handicap, pendant le temps scolaire. La plupart des écrans d'ordinateur, de tablette ou de téléphone émettent une lumière enrichie en bleu. Chez l'homme, la lumière bleue a des effets physiologiques et des risques associés spécifiques, à savoir, principalement, une atteinte de la rétine, d'une part, et une perturbation de l'horloge biologique, d'autre part. L'exposition à la lumière bleue pourrait notamment être un des facteurs à l'origine de pathologies rétiniennes, telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les jeunes constituent la population la plus vulnérable, car leur exposition cumulée au cours du temps sera plus importante et leur cristallin transparent ne filtre pas la lumière bleue : en vieillissant, le cristallin s'opacifie et prend progressivement une coloration jaune, faisant office de filtre physiologique.

Merci,